La séance est ouverte le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 13 janvier a été publié sur le site internet du Sénat il y a-t-il des observations, je n'en vois pas le procès-verbal est donc adopté, chers collègues, nous allons passer à la séance des questions orales, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Sabine Van Egg au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. La parole est à notre collègue. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention de monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'alimentation sur la problématique des établissements d'abattage non agréés les E. A. en effet aujourd'hui les exploitations agricoles qui élève des volailles palmipèdes gras et des lapins sont en droit d'avoir des ENA sur leur exploitation pour abattre découpé et transformer les animaux élevés sur place, la direction générale de l'alimentation estime à 2700 le nombre de ces ateliers, en France, l'essentiel des produits issus de ces ateliers sont commercialisés en circuit court et de proximité circuit plébiscité, notamment depuis la crise sanitaire de plus, un atelier d'abattage découpe et transforme et embauche à lui seul un à 3 ETP, c'est le règlement européen 853 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale qui permet à ces établissements d'exister, de découper les produits dans un cadre très strict, le règlement d'application 2000 1785 de la Commission européenne complète le règlement 853 2004 et étant la dérogation à la transformation dans ses ateliers dérogations temporaires qui se termine fin de cette année la suppression éventuelle de ce droit, aurait des conséquences très négatives pour les exploitations concernées, en effet, la transformation des produits est un élément clé dans l'équilibre économique des ateliers, des exploitations, les éleveurs transformant leur viande non pas les capacités matérielles et financières d'investir dans un abattoir agréé, ce qui pénaliserait fortement l'économie locale freinerait le développement des circuits courts et pourraient faire disparaître à terme, de nombreux savoir-faire et employes, je souhaite donc savoir ce que le gouvernement entend faire afin de garantir la pérennité des ateliers concernés des exploitations qui les ont développées afin de répondre à la demande sociétale croissante en produits locaux vendus en circuit court et respectant le bien-être des animaux, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Julien de Normandie Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci beaucoup, madame la présidente, messieurs et mesdames les les sénateurs et sénatrices madame la sénatrice Sabine Van Egg, vous l'avez dit, ces établissements d'abattage non agréés, les femmes à ENA sont des outils extrêmement important pour notre territoire, il y en a près de 3000. ce sont aujourd'hui des lieux sur lesquels repose notamment les circuits courts, il faut que mais c'est mon attachement à la promotion des produits frais, des produits locaux, j'allais dire d'ailleurs votre attention et celle de vos collègues sur la plateforme nationale que nous avons lancé il y a 15 jours, qui s'appelle frais et local point fr qui permet à tous nos concitoyens de repérer autour de chez eux, là ou des ventes directes sont possibles, des ventes à la ferme des fantômes, producteur et donc les oeufs à asthme des éléments essentiels et c'est vrai que le règlement européen prenait fin au 31 décembre 2020, ce règlement européen ne permettait plus

de prolonger la vente de viande fraîche, mais pas de viande transformée, ce qui est absolument ubuesque, dès lors que ces ENA permettent par là même de faire une première transformation des produits carnés qu'le mettent à disposition ensuite des consommateurs on s'est beaucoup mobilisé le gouvernement moi-même j'ai à plusieurs plusieurs reprises pardon porté ce sujet ou au sein de l'enseigne l'enceinte du conseil des ministres européens, j'en ai parlé à plusieurs reprises à la commissaire européenne en charge de ce dossier Madame Stella Kyriakides

de continuer à fonctionner, je vous détaillerait tout cela par écrit pour que un écrit puissent également être fait sur le sujet, mais c'était pour moi très important que la poursuite des et a soit possible et ces choses qui est fait puisque nous avons trouvé une solution : le permettant, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, chers collègues, vous avez 30 secondes pour répliquer. Oui, merci Monsieur le Ministre, je viens bien entendu ce que vous venez de dire je compte bien sûr sur votre intervention et mes collègues, je ne dis pas qu'il partage mon sentiment ici et je vous le répète, Monsieur le Ministre, pensions aux petits éleveurs qui se trouveraient encore une fois, pénaliser face aux plus puissants, et avec eux toute une frange de l'économie locale, je vous remercie. l'alimentation. La présidente, monsieur le ministre, le 9 novembre dernier la Commission européenne a décidé de prendre des sanctions douanières contre les États-Unis, ces mesures impliquent notamment une surtaxe sur les produits agricoles et agroalimentaires, or la noix comme d'autres fruits à coque une s'y trouve pas la production de noix en France s'élève en moyenne à 40000 tonnes par an, dont 20000 tonnes en région Auvergne-Rhône-Alpes parmi cette production régionale, la noix de Grenoble Appellation d'Origine protégée à laquelle vous imaginez que je suis très attaché fait office de locomotive en tirant toute la filière vers le haut, la production de cette loi au pays représentent environ 12 à 14000 tonnes par an et une majorité environ 60 % est exportée chaque année vers l'Europe, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne étant les principaux clients, or sur le marché européen, la concurrence est très forte, les États-Unis, ils n'ont, en effet, les marchés, avec une production qui avoisinerait en 2020, le 800000 tonnes pour le volume comme pour les tarifs, la France n'est pas en mesure de rivaliser avec cette force de frappe, il est bien entendu que les modes de production diverge largement entre le système californien ultra-productiviste et notre système traditionnel français qui fait la renommée de notre agriculture toute entière dans sa décision, la Commission européenne a pourtant ignoré les noix et la plupart des fruits à coques qui sont exclus de la surtaxation, or si l'objectif de cette mesure et de faire pression sur les États-Unis, les fruits à coque pourrait être un levier efficace, en effet, l'Europe est un des premiers clients des États-Unis, tant pour la noix en coque que pour le CERN ou intégrer les noix, dans ces mesures permettraient donc aux producteurs français de redevenir concurrentiel sur le marché européen, l'enjeu n'est rien de moins que la protection des productions hexagonales et de notre agriculture, dans ce cas-là de qualitative et de singulières aussi, monsieur le ministre comment la France pourrait-elle intervenir auprès de la Commission européenne afin qu'un élargissement du produit concerné par la taxe sur taxation puisse intégrer les noix et les fruits à coque qui qui en sont aujourd'hui exclus, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le, le sénateur Didier Rambaud d'abord je voudrais saluer tout le travail qui le voteront en soutien de la filière noix noix de Grenoble mais mais d'autres types de de production locale, je connais votre attachement à ce sujet, toute l'action que vous menez, on en parle régulièrement la question que vous posez, c'est : comment fait-on pour. Augmenter la production, et singulièrement de la consommation des des noix dans notre beau pays, avec la pression de l'importation de noix de pays extérieurs et à ce titre vous proposer d'utiliser le le contentieux que nous avons en ce moment entre l'Union européenne et les États-Unis lié au contentieux Airbus-Boeing pour faire en sorte que des pressions avec des barrières tarifaires douanières en terme de mesures de rétorsion soient mises en place contre l'importation des fruits à coque et notamment des Noirs des États-Unis, je comprends l'idée tout tout sujet doit être regardée et je m'y engage, ceci étant étant dit je, je, l'objectif du gouvernement c'est de réussir. Sans faire preuve d'aucune naïveté, c'est pour ça qu'on a mis des mesures de rétorsion et que la France avait poussé par ces mesures de rétorsion au niveau européen mais d'aboutir à une désescalade avec la nouvelle administration Biden et à l'atterrissage d'un compromis sur ce contentieux Boeing Airbus ce contentieux, il fait des victimes collatérales français toute la filière du vent qui, vous le savez, profondément impacté par les mesures prises par les États-Unis et je sais que la présidente, il est assez sensible et donc notre objectif c'est désescalade et ne surtout pas faire de ces sanctions, quelque chose de pérenne et donc je ne pense pas que ce soit le bon vecteur pour asseoir sur la durée de la production des fruits à coque en France, je pense qu'en revanche, si vous l'avez dit-il, une autre question qui se pose, mais qui va être un combat de longue haleine mais que je voudrais porter moi lorsque j'aurai la présidence du Conseil européen des ministres de l'agriculture si vous savez le fameux article le fameux article 44 de la loi Egalim qui avait été modifié dans le projet de loi portant sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour la betterave, 10 ans, est ce que on ne devrait pas regarder le mode de production culturelle quand on permet l'importation d'un certain nombre de produits dès lors que ces modes de production culturelle ne respecte pas les principes de base, notamment environnementaux qui régissent le marché commun et je suis prêt à travailler avec vous sur ce sujet, la question de la loi, il y a, qui sont la noisette, également, c'est quelque chose qu'on a pu utiliser par exemple sur un certain nombre d'importation de cerises depuis la Turquie et donc regardons cela en somme, c'est un vrai vrai combat au niveau européen qui prendra du temps et je pense que cette question doit être posée, c'est un vrai sujet politique. Merci cher Ministre vous avez 30 secondes, si vous souhaitez répondre chers collègues. Merci monsieur le ministre pour la la clarté de vos propos, une fois de plus, et puis surtout pour les les perspectives que que vous tracez et puis comme vous, je place beaucoup d'espoir aussi, avec l'arrivée de l'administration by donne qui j'espère va réparer un petit peu la la paix commerciale entre les États-Unis et et l'Europe, sans être pour autant être naïf quant à leur protocole protectionnisme dont ils font toujours preuve merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de notre collègue sénateur Jean-François Rapin au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite aujourd'hui, Monsieur le Ministre vous interpeller sur les moyens alloués aux agriculteurs français pour répondre aux nouvelles exigences climatiques comme le soulignait un rapport sénatorial sur la résilience agricole et alimentaire, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la voie d'une production plus respectueuse de l'environnement, afin de les inciter davantage les politiques publiques actuelles agissent par la contrainte en durcissant les normes applicables aux paysans, au détriment de leur compétitivité, les travaux de mon collègue Laurent Duplomb dresse le constat selon lequel le respect de ses objectifs réduit d'autant plus notre capacité productive agricole au point que l'on risque de perdre notre excédent dès 2023. Dans le même temps des pays dont le modèle agricole, hé bien moins respectueux de ces normes continueront d'exporter leur production vers la France, notamment pour répondre à l'injonction des prix bas, étouffant ainsi les agriculteurs français, on voit déjà d'ailleurs poindre un débat entre producteurs et grande et et grands outils de de distribution face à cette situation, la recherche scientifique et technologique, peinent à trouver les moyens suffisants pour avancer dans une direction qui permettrait de restaurer notre puissance puissance productive sans dégrader les écosystèmes et en s'adaptant au changement climatique, comment le gouvernement envisage-t-il d'améliorer l'accompagnement des agriculteurs, mais aussi des acteurs de la recherche afin de permette de trouver une conciliation entre le respect des exigences climatiques et notre souveraineté agricole, quel en serait le calendrier d'action, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'agriculture, de l'alimentation. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs monsieur le le sénateur Jean-François Rapin, la question que vous posez, elle est essentielle, j'ai déjà eu l'occasion de de l'évoquer ici et j'lu les travaux faits par le Sénat et singulièrement par le sénateur Laurent Duplomb sur ce sujet, la base de l'agriculture de l'agronomie, c'est l'eau. On peut prendre le sujet par tous les bouts, on peut avoir un certain nombre de prophète qui consiste à dire qu'il sera possible demain de faire de l'agriculture sans eau, tout ça n'est pas vrai : la base de l'agriculture, c'est l'eau aujourd'hui il nous faut absolument affronter ce sujet avec beaucoup de de détermination, il faut le faire aussi sereinement parce que depuis que l'homme est sédentaire, le conflit d'usage de l'eau existe c'est vrai depuis des millénaires, et donc, face à ça, il faut se dire que la première chose pour se prémunir contre les aléas du changement climatique, c'est d'améliorer la gestion en nous, dans notre pays, c'est un des objets du plan de relance, c'est un des objets de mode projet que j'ai mis en place au sein du ministère de l'agriculture, on a identifié territoire après territoire : tous les projets d'eau pour voir quels sont les accompagnements à porter toujours dans la concertation avec les fameux projets territoriaux de gestion en haut qui aujourd'hui maille le territoire mais à la fin décembre pour faire sortir ces projets qu'on ne concertation dure 8 à 10 ans c'est qu'à la fin, c'est une mauvaise concertation une concertation importante, elle doit être canalisée dans le temps, sinon à la fin tout le monde s'épuise, donc la première chose c'est d'affronter la question de la gestion de l'eau, la 2ème chose c'est d'accompagner nos agriculteurs dans des investissements de protection là où l'eau, c'est la prévention dans la protection dans le cas du plan de relance, on a mis en place une ligne de 100 millions d'euros pour financer des équipements de lutte contre les aléas du changement climatique, systèmes d'irrigation individualisé, système de performances, système de filets anti-grêle etc etc etc, les lignes sont ouvertes les dossiers commencent à affluer la 3ème prend le 3ème point pardon sur cette question de la souveraineté agricole ça fait quoi, ce que je disais à votre collègue Didier Rambaud tout à l'heure et puis le 4ème point est le sujet de la recherche pas si vous avez vu sur des débats enflammés du fait de mes prises de position sur ce qu'on appelle l'embêter sur Les MDT, typiquement, vous avez d'illustres scientifiques qui vous disent que ça peut être une aussi une solution pour déterminer comment trouver des plantes qui soient plus résilientes vis-à-vis de ces changements, les embêter, c'est une pratique, c'est en gros une accélération de la sélection variétale, c'est-à-dire qu'en gros, ça permet de déterminer aujourd'hui une plainte qui probablement serait de manière naturelle, intervenu à un moment donné, dans un lieu donné de façon naturelle, sauf que vous accélérer cette sélection variétale voilà, vous voyez mon approche très pragmatique sur ce sujet, ce qui est sûr, c'est que la mère des batailles, c'est celle-là, il n'y a pas d'agriculture possible sans une gestion efficace en haut et sans une recherche sur la résilience de de nos plantes pour pouvoir affronter les épisodes de sécheresse, les uns après les autres et de manière générale, le réchauffement climatique, ce que je dis là pour les pentes, c'est tout à fait vrai aussi pour les arbre et la forêt quand vous prenez une très belle et très aujourd'hui dans notre pays, qui subissent le changement climatique, la même réflexion doit être apportée, y compris dans nos massifs forestiers. Merci monsieur le ministre, chers collègues, il vous reste un peu plus d'une minute pour répliquer. Monsieur le Ministre, merci de votre réponse, bien sûr que j'ai vu dans le budget 2021, les propositions qui ont été faites et et j'espère qui qui se qui s'acteurs ont officiellement, néanmoins, nous sommes toujours demandeur d'de plus d'argent et dans les situations. On connaît actuellement, c'est difficile, la question est, à mon avis, celle des priorités est ce qu'on fait aujourd'hui de son de cette échéance climatiques une priorité en terme de recherche et de développement, agroalimentaire, si c'est une priorité, dont acte, et à ce moment-là on on met les moyens, la 2ème question que je voulais évoquer avec vous, c'est celle des prix, je l'ai dit dans mon propos, on voit la bataille des prix entre producteurs et distributeurs recommencer et prendre une ampleur peut-être comme jamais avec des mots qui sont dits et qui sont, aujourd'hui, je trouve très violent, est, il est temps aussi de permettre aux agriculteurs au travers cette recherche d'avoir des coûts de production qui restent compétitifs pour permettre à la grande distribution effectivement de satisfaire le pouvoir d'achat des consommateurs, je vous remercie. Merci l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Hélène Conway Mouret au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe, des affaires étrangères chargée du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, merci, cher collègue. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaite vous alerter par cette question sur la situation financière des établissements de la Mission laïque française au Liban, la situation politique, économique, sociale de ce pays et critique : elle s'aggrave, malheureusement avec la pandémie et l'explosion un ou 2020, qui a dévasté le quartier du port de Beyrouth, nous a fait prendre prendre conscience du soutien dont a besoin ce pays ami, nous y avons répondu en envoyant au Liban une aide humanitaire d'urgence avec plusieurs tonnes de matériel sanitaire, nous avons également apporter un soutien financier de quelque 50 millions d'euros pour la santé, l'emploi, le logement, la culture, l'éducation, enfin, nous avons attribué 20 millions d'euros pour venir en aide aux réseaux des 50 écoles francophones, dont 4,4 millions d'euros en faveur de 5 établissements de la Mission laïque française, je ne peux que saluer ce soutien en faveur de l'enseignement français dans ce pays francophones et francophiles, malheureusement, il semblerait que ces crédits ne soient pas suffisants, en effet, les 5 lycées la Mission laïque avec leurs 7100 élèves sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique locale, le pire est sans doute à venir avec un déficit cumulé estimé à 10 millions d'euros au moins si rien n'est fait pour les aider, MLF ne peut pas compenser, seul ce déficit, je souhaiterais savoir si les aides attribuées en 2020 sera reconduite cette année pour aider ces 5 établissements de la Mission laïque à traverser cette crise et éviter leur fermeture. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. La présidente, madame la sénatrice, je partage votre préoccupation sur la situation au Liban qui connaît aujourd'hui une crise multiple profonde à la fois économique, social, politique et sanitaire cette préoccupation, vous le savez, celle portée par le prion de la République, qui s'est rendu au Liban, à 2 reprises depuis l'explosion dans le port de Beyrouth cet été et dans ce contexte difficile, nous portons évidemment une attention toute particulière, vous l'avez rappelé la situation, les 55 établissements de l'enseignement français au Liban, qui est le 1er réseau au monde par le nombre d'élèves scolarisés, près de 60000 à la dernière rentrée, dont une majorité d'ailleurs d'enfants libanais parmi ces établissements, 5 sont gérés directement par la Mission laïque et 5 autres y sont affiliés, tous ont été affectées par cette crise économique par la crise sanitaire et par les destructions liées aux explosions du début du mois d'août dans le port de Beyrouth, c'est pourquoi nous avons veillé à ce que ces difficultés particulières soient bien prises en compte, vous l'avez rappelé dans le cadre du plan de soutien du réseau d'enseignement français à l'étranger, préparé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et les établissements français au Liban, ont reçu, en effet, un peu plus le 20 millions d'euros, dont 7 millions pour l'aide à la reconstruction, ce qui a fait du Liban le 1er bénéficiaire de ce plan d'aide et cela est bien légitime parmi les 5 établissements que j'évoquais de la Mission laïque française, un effort important a été fait, vous l'avez également souligné avec 4,3 millions d'aides budgétaires attribués je souligne que 2 de ses établissements ont reçu en particulier plus de 800000 euros chacun, ce qui représente au total pour ces 5 établissements 20 % des crédits de soutien destiné aux réseaux libanais des établissements conventionnés de la Mission laïque française au Liban ont pu compter aussi sur un soutien important de la part de l'État et puisque vous posiez la question du la prolongation de ce soutien, je souligne que le déploiement de ces aides, engagé en 2020, va se poursuivre sur le 1er semestre 2021 au total, la Mission laïque française dans d'ailleurs a reçu plus de 10 millions d'euros d'aide pour l'ensemble de son réseau d'établissements dans le monde, là aussi, c'est environ 20 % du plan global débloqués pour notre réseau à l'étranger, madame la sénatrice en 2021 comme en 2020, vous y fait écho, nous resterons mobilisés auprès des familles et des établissements scolaires du Liban avec une aide significative dont le versement se prolongera et bien sûr, nous resterons vigilants pour, le cas échéant, adapter ou renforcer le soutien nécessaire, nous ne laisserons pas tomber notre réseau en général et ce réseau exceptionnel que nous avons, au Liban, en particulier. Merci monsieur le secrétaire d'État, la parole est à Madame Hélène Conway Mouret pour un peu plus d'une minute. merci monsieur le ministre, alors je crois que vous avez très justement rappelé comme je l'ai fait moi-même ce que nous avons fait ce qui m'intéresse, par cette question, c'est ce que nous allons faire allons-nous continuer à aider ces établissements scolaires pour rassurer les familles qui font de gros efforts qui font de gros sacrifices pour scolariser leurs enfants dans des établissements où les frais d'inscription, enfin les frais écolage sont quand même élevés mais également pour tous les personnels qui travaillent dans ces établissements, parce que, aujourd'hui, la situation est est vraiment très très critique dans ce pays, j'ai noté, il y a quelques jours, ce que le quotidien Al-Akhbar titrait il disait : c'est l'enfer, pas simplement de regarder ce que nous avons fait et nous en réjouir, je crois que c'est le cas, mais ce que nous allons faire, vous parlez d'un prolongement du soutien, ce que j'aurais aimé avoir de votre part mais peut-être que nous pourrons l'avoir par écrit, si je ne l'ai pas eu oralement, ce matin, c'est exactement en quoi va va constituer ce ce ce soutien prolongement de des des crédits votés l'année dernière, c'est très bien mais qu'allons-nous apporter en crédits supplémentaires,

Merci madame la présidente, monsieur le Ministre. Un bulletin de vote et plus fort qu'une balle de fusil cette citation et d'Abraham Lincoln et elle nous interpelle évidemment sur le rôle de la démocratie. Le taux de participation chez les Français de l'étranger il pour le comprendre, il dépend du fait que beaucoup de Français de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parcourt des centaines de kilomètres pour aller mettre leur bulletin de vote, le temps d'une élection je vais, je souhaite vous interpeller sur 3 points relatifs à la participation électorale des Français de l'étranger, le 1er point c'est la nécessité de mettre à jour la liste des bureaux de vote et d'avoir une liste des bureaux de vote, la plus importante possible, pourquoi, parce que pour par exemple établir une procuration, souvent on attend une tournée consulaire, c'est-à-dire des agents qui se rendent dans la commune où on de résidence, or avec la crise pandémique évidemment la mobilité est contrainte et lors des élections européennes l'année dernière, enfin, lors des dernières élections européennes, par exemple, je sais, c'est, c'est un exemple parmi d'autres, mais le bureau de vote d'Al-Khobar qui se situe à 420 kilomètres de Ryad 420 c'est-à-dire pour aller voter,

revu 2ème élément, le vote par correspondance, il y a 2 2 éléments dans le vote par correspondance, le vote par correspondance électronique le vote par Internet. Mais également dans un certain nombre de pays où la Poste fonctionne parfaitement bien. le souhait du rétablissement et je l'avais notamment défendu dans un amendement du rétablissement du vote par correspondance papier quant à la Poste donne parfaitement satisfaction, c'est également un moyen de permettre aux Français de l'étranger de participer. Et enfin 3ème élément, c'est plutôt une proposition nouvelle, que je souhaite, maître sur la table et pour laquelle je souhaite interpeller le gouvernement. Parmi les électeurs français, qu'il soit en métropole dans les Outre-Mer les seuls Français qui ne disposent pas de carte d'électeur de carte électorale cette carte tamponnée au moment du vote dans un bureau de vote, ce sont nos compatriotes qui vivent à l'étranger, et donc je soumet l'idée de créer une carte d'électeur pour les Français de l'étranger, qui a un très fort, un fort caractère symbolique d'appartenance à la citoyenneté, citoyenneté, tout comme elle est remise, cette carte d'électeur, lors de la cérémonie d'accueil à la nationalité française ou pour les jeunes majeurs et enfin cette carte d'électeur pourrait être dématérialisé et imprimé par les Français eux-mêmes, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Madame la présidente, monsieur le sénateur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'attache en effet à faciliter et encourager comme vous y avez rappelé votre attachement, la participation aux élections de nos ressortissants vivant à l'étranger, ce sera notamment le cas pour les prochaines élections consulaires, prévu les 29 et 30 mai prochain pour lesquelles mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne est engagée pour organiser plusieurs campagnes de communication particulier afin d'informer les électeurs sur les modalités de ce scrutin, comme sur le rôle des conseillers des Français de l'étranger. S'agissant de la dernière proposition formulée d'une proposition de 2 cartes électorales qui serait destiné aux Français de l'étranger, d'abord je veux rappeler l'existant, la présentation d'une pièce d'identité française ou une carte d'inscription au consulat qui peut vous le savez, de s'être imprimé directement par l'usager fait aussi office de démarche civique suffit aujourd'hui aux opérations électorales il y a l'impératif d'efficacité, de rapidité qui je crois est remplie, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à ce stade de donner suite à l'idée que vous soumettez à nouveau ce matin de carte électorale pour ajouter un document possible à ces formalités existantes mais je suis presque avec Jean-Baptiste Lemoyne, nous regardions sur le point que vous soulignez, c'est-à-dire comment mobiliser, informer mieux nos concitoyens par exemple par des courriers électroniques où ce type d'instrument, j'en ferai part à Jean-Baptiste Lemoyne, pour qu'on continue avec vous cette réflexion s'agissant des bureaux de vote, nous avions prévu en mai 2020, un dispositif très étendue 464 bureaux de vote sur 358 6, ce qui représente déjà un effort de mobilisation important pour mai 2021, le dispositif doit naturellement tenir compte, vous le comprendrez, avec les incertitudes qui s'y attachent, de la situation sanitaire, mais nous ferons en sorte évidemment d'avoir une couverture une accessibilité la plus large possible, nous travaillons avec nos postes diplomatiques et consulaires pour adapter définir ce dispositif dans ce contexte, avec évidemment 2 impératifs qui sont le même garantir la sécurité sanitaire des électeurs garantir aussi la sécurité sanitaire des volontaires et des agents qui tiendront ses bureaux cet impératif est essentielle et sur l'idée d'une liste à jour, nous y travaillons, bien sûr, pour informer au mieux s'agissant enfin du vote par correspondance sur le vote électronique, nous n'avons aucun doute, c'est un système simple et sûr, vous l'avez rappelé dont on doit encore mieux faire connaître l'existence nous avons, je le dis sincèrement plus de réserves sur le système de vente le vote par correspondance postale parce que vous avez cité les cas où cela fonctionne bien, il y a aussi beaucoup de pays où il y a une fiabilité aléatoire, très imparfaite de la circulation de la transmission postal et à risque aussi, et cela vaut en revanche pour tous les pays de contentieux électoraux qui sont importants, mais je suis prêt, là encore, à ce qu'avec Jean-Baptiste Lemoyne, peut-être dans un souci de différenciation accrue que vous évoquiez, nous continuerons avec vous cette réflexion mais je tenais à vous faire part de ses réflexions de manière transparente ce matin. la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la mise en oeuvre et concrète du plan de relance, et plus particulièrement sur les possibilités de financer des projets structurants sur le département du Gard la crise sanitaire que nous traversons aura d'importantes répercussions sur notre économie, dans beaucoup de secteurs, ses conséquences économiques se font déjà ressentir dans ce contexte d'annonce d'un plan de relance, doté de 5 milliards d'euros, est une bonne nouvelle pour l'activité des entreprises pour l'emploi dans beaucoup de départements, il existe des projets structurants fortement inspirée par les habitants, certains d'entre eux sont évoqués, attendu avec impatience depuis maintenant plusieurs décennies non seulement ces projets sont attendus, mais il faut souligner que, compte tenu, impossibilité des collectivités territoriales, de les financer, où il s'est souvent difficile de dégager des financements pour ces investissements s'est installé, il y avait des conséquences économiques et sociales que nous connaissons dans le Gard, le 2ème, département le plus industrialisé cette grande région d'Occitanie avec quelques fleurons comme SNR Berlin gérée, Royal Canin, mais il n'en demeure pas moins qu'il est le 4ème, département le plus pauvre de France, ce n'est pas une fatalité, nous avons besoin d'infrastructures modernes durables et efficaces, songez que la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 106 entre Nîmes et Alès de grandes villes distantes d'une quarantaine de km une préfecture une sous-préfecture de bassins d'emplois industriels et tertiaires débuté par la mise en place d'un chantier de ce 1er tronçon en 1998 n'est toujours pas achevé, heureusement, monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, nous avons pu bénéficier de fonds structurels européens, à l'époque pour financer ses projets, le Gard, a d'ailleurs toujours été l'un des départements les plus performance pour obtenir des subventions de l'Europe, je profite de votre présence pour émettre le souhait que dans le cadre d'un nouveau projet de budget européen pur annuel 2021 2027 que le Gard puisse continuer à bénéficier, ce sont donc, monsieur le ministre, 8 petits qui sont des chefs nécessaires pour achever la liaison entre Nîmes RDS préalablement au contournement ouest de Nîmes la maîtrise d'ouvrage est porté par l'État, je ne doute pas que le gouvernement aura à coeur d'en faire l'une des priorités du plan de relance ses campagnes le contournement ouest et sans barreaux verra enfin le jour très prochainement, je reviendrai vers vous également pour évoquer d'autres projets, notamment la rocade nord du du du département du Gard, porté par le conseil départemental dont j'ai été le président pendant plus de 5 ans qui permettra un accès Direct à la gare TGV de Nîmes Pont du

pour permettre non seulement dans le département de rebondir rapidement à la sortie de la crise sanitaire, mais également pour envisager un futur développement économique durable au service de notre population, merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes pour 2 minutes 30, s'il vous plaît. à la présidente, monsieur le sénateur vous interrogez le gouvernement et. Plus particulièrement ma collègue ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au sujet de la mise en oeuvre du plan de relance et de ses répercussions en particulier sur le projet du contournement ouest de l'île, combien d'abord de rappeler que le plan de relance français financés, cela me tient à coeur à 40 % par le plan de relance européen s'articule autour de 3 axes, comme vous le savez, l'écologie et la compétitivité et la cohésion notamment des territoires et dans ce cadre et un certain nombre, c'est vrai, d'opérations relatives relatives au réseau routier national inscrite au contrat de plan État-Région pourraient bénéficier d'un financement permettant une accélération de leur mise en oeuvre, mais je le souligne de manière très l'effort de relance qui s'étale sur la période 2021 2022 conduit à privilégier, dans ce cas, de les opérations qui peuvent être engagées d'ici 2022 le contournement ouest de Nîmes bénéficient, vous le savez, d'une inscription d'ores et déjà de 8,3 millions contrat de plan État-Région. Qui se termine 2015, 2020 afin de mener les études et de procéder aussi plus concrètement aux acquisitions foncières, le financement des travaux n'est pas encore bouclé, à ce jour et le déroulement des études comme les procédures ne permettent pas aujourd'hui d'envisager le début des travaux effectifs avant l'année 2022, c'est à ce titre que dans le cadre spécifique du plan de relance à ce stade, cette opération ne nous paraît pas éligible, mais l'État travaille néanmoins à la à la finalisation des études préalables du contournement ouest de Nîmes dans la perspective de soumettre le projet à l'enquête publique préalable à cette déclaration d'utilité publique au 1er semestre de l'année prochaine et en particulier la possibilité d'intégrer une liaison entre le contournement ouest et la RN 113 qui est une demande forte que vous portez et que portent les élus des collectivités locales est en cours d'étude comme vous le savez, donc l'année 2021 doit être utile, consacrée à la consultation des collectivités territoriales concernées et des services de l'État sur le projet modifié afin de prendre en compte les remarques émises lors de la concertation, de 2017 qui avait précédé la saisine de l'autorité environnementale pour avis sur l'évaluation environnementale du projet en tout état de cause, la question du financement, les travaux du contournement ouest trouvera sa place lors des négociations de la prochaine programmation financière contrat de plan État à partir de 2023 pour son financement de travaux effectifs le volontarisme financier de l'État et des collectivités territoriales serait alors déterminant pour la poursuite de ce projet, je souligne aussi la bonne prise en compte du du de d'autres projets d'infrastructures modernes et sûrs, comme vous l'avez dit, la rocade nord en particulier et je m'engage il travailler si vous le souhaitez, avec vous, pour prolonger cet échange sur le financement des financements européens additionnels qui pourraient sur ses projets d'infrastructures et aider à leur accélération et à leur réalisation. Merci monsieur le secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle maintenant la question orale du président Jean-François Longeot au ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la situation dans le département du Doubs et plus particulièrement dans l'agglomération de Montbéliard où les habitants, les services de police et de secours subissent régulièrement des violences, des incendies et des saccages de l'espace public, or malgré des échéances des échanges avec la préfecture, la venue ponctuel de renforts de compagnies républicaines de sécurité, aucune amélioration n'apparaît, bien au contraire, la situation se dégrade escalade de la violence est bien réelle, montrant l'inefficacité de la politique de sécurité publique menée sur les territoires aujourd'hui les services de secours et de sécurité ne peuvent intervenir sereinement par manque de directives courageuse d'intervention et de rétablissement de l'État de droit, dans chacun de ces quartiers, les habitants sont en danger et subissent chaque jour des dégradations et des violences aussi, dans ces conditions, je tenais tout d'abord à remercier le ministre pour son écoute lors d'une rencontre organisée au ministère de l'Intérieur en décembre dernier et souhaité de surcroît connaître vos intentions pour rétablir l'ordre au public et la suite sécurité sur ce site, sur ce territoire nord Franche-Comté, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, en matière de sécurité, vous l'avez rappelé les attentes des Français sont fortes, et le gouvernement, vous le savez est pleinement mobilisé pour y répondre à cette mobilisation, c'est d'abord celle des policiers et des gendarmes sur le terrain et c'est pourquoi nous avons décidé de renforcer leurs moyens, le plan de relance se traduit par exemple par une augmentation du budget de 325 millions d'euros pour la police nationale et ce sont 10000 policiers et gendarmes supplémentaires qui sont recrutés d'ici à la fin du quinquennat pour renforcer les effectifs là où les besoins sont de se par ailleurs après les pistes ambitieuse tracé par le Livre blanc de la sécurité intérieure, dont certaines d'ailleurs se concrétise avec par exemple l'expérimentation de direction départementale de la police nationale, le bobo de la sécurité annoncé par le président de la République en décembre et qui sera annoncé le 25 janvier va constituer une nouvelle étape avec les forces de l'ordre des maires, des parlementaires, nous allons identifier les nouveaux moyens dont il nous faut doter à court terme, les policiers et les gendarmes et à plus long terme bâtir ensemble les bases d'une nouvelle loi de programmation que nos forces mérite et que vous avez appelé de vos voeux, ressens maintenant à votre département, Monsieur le Sénateur, nous connaissons vos préoccupations et les cabinets du ministère de l'Intérieur, ont eu l'occasion de recevoir les élus locaux début décembre et, en 1er lieu je voulais vous assurer, au nom du ministre de l'Intérieur, que nous ne laisserons rien passer en la matière, nous intervenons chaque fois que l'ordre public est contesté les violences, les désordres à Montbéliard, comme ailleurs, les attaques contre les policiers contre tous les représentants d'institutions publiques sont particulièrement inadmissibles et à Montbéliard, comme ailleurs, vous savez que nos policiers sont pleinement mobilisés et je note, même si cela ne saurait évidemment minimiser les problèmes qui existent que plusieurs indicateurs témoignent de l'efficacité de leur travail dans le département, par exemple, une baisse de 13 % des violences aux personnes, et de près de 18 % des atteintes aux biens, en 2020 dans la circonscription de police de Montbéliard et Héricourt la prochaine arrivée de 8 nouveaux gardiens de la paix supplémentaires va permettre, nous l'espérons, de poursuivre cet effort qui constaté depuis l'été dernier,

je crois que cette période que vous avez évoquée, elle a permis aux forces locales de faire avancer l'enquête, notamment le 2 décembre, soit 10 jours après les faits qui ont été évoqués, 2 individus ont été interpellés depuis les violences urbaines ont baissé d'intensité et sont même devenues quasiment inexistantes dans le quartier, cité 16 faits de violence urbaine dont quatre dans ce quartier ont seulement été enregistrés dans la circonscription en décembre et quatre seulement, entre guillemets, et aucun dans la zone de sécurité prioritaire je redis parce que ça peut paraître anecdotique mais en novembre était recensé 29 faits de violence urbaine dans la CIA IST Montbéliard Héricourt, dont 9 ans ZSP donc on voit qu'il y a véritablement une baisse à Montbéliard, comme partout ailleurs, monsieur le sénateur, je voudrais vous assurer du soutien total de l'État du ministre de l'Intérieur et moi-même pour être avec vous au côté des élus locaux et je voudrais terminer en saluant à cet égard l'engagement de la municipalité et des élus en faveur de la sécurité parce que je crois que c'est ensemble que nous pouvons garantir aux Français à la sécurité et la tranquillité qu'ils attendent légitimement dans leur vie quotidienne, je crois que ce travail partenarial il doit véritablement être salué, je vous remercie. Je rappelle que vous avez 2 minutes 30 de temps de parole pour les autres réponses qui sont à à venir, merci madame la ministre, chers collègues, il vous reste une minute, un peu plus d'une minute pour répliquer si vous le souhaitez. merci, Madame la Ministre, pour vous, pour votre réponse et merci effectivement pour l'entretien que nous avons eu au ministère de l'Intérieur, j'étais avec ma collègue : Annick Jacquemet effectivement présents à cette rencontre je crois que ce qui s'est passé à la Petite Hollande c'est un c'est un quartier de de de Montbéliard où il fait bon vivre mais aujourd'hui c'est très compliqué pour pour les populations qui habitent dans ce quartier depuis des années et qui aimeraient avoir un peu de tranquillité il faut qu'il y a une vraie relation entre entre votre ministère et celui de la justice, hein, parce que il y a trop de laxisme à l'égard de ces personnes, il est quand même inadmissible qu'avec un engin de chantier, on aille faire tomber des candélabres, sur lesquels la municipalité, 3 jours avant, avait installé des caméras de surveillance, je crois que c'est, c'est quelque chose d'intolérable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre et je crois qu'il faut qu'il y ait cette véritable relation entre votre ministère, ceux du ministère de la justice, parce que ce sont des actes effectivement non seulement qu'il faut condamner, mais qu'il faut punir, merci. Merci, cher collègue lors du jour appelle la question orale de notre collègue sénateur Daniel Laurent au ministre de l'Intérieur. Oui, madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur la défense extérieure contre l'incendie qui, depuis la réforme de 2015 ne répond plus à une norme nationale mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet en concertation avec les collectivités territoriales si la sécurité des habitants est une priorité pour les élus l'interprétation souvent très stricte des dispositions des règlements départementaux conduit à des contraintes disproportionnées sur certains territoires et à des coûts de mise aux normes très important sur les Budgets pour les Budgets communaux en Charente-Maritime, grâce à la mobilisation des élus, la DETR et prioriser pour les dossiers de mise en conformité le département apporte également sa contribution dans la limite des plafonds d'intervention légaux, ce sont des décisions importantes pour alléger la facture des communes mais pour très déficitaire, elles devront étaler la mise en conformité sur plusieurs années dans le cadre des schémas communaux communaux de défense extérieure contre l'incendie, obérant ainsi le développement d'autres projets et la dynamique de nos territoires ainsi de nombreux permis de construire sont refusés en raison de l'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation dans une décision du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers fait état que le règlement départemental de défense contre l'incendie qui relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ne saurait être opposable aux demandes d'autorisations d'urbanisme cette jury prudence a permis de débloquer des dossiers, quand bien même les communes ne seraient pas mises en conformité avec le règlement départemental, toutefois, il convient de lever toute insécurité juridique comme nous le demandent les élus à ce jour, aucune compagnie d'assurance ne suis retourné contre un maire ou une commune mais il convient de prévenir ce risque, en cas d'incendie d'une construction situé dans une zone ne répondant pas aux critères de règlement départemental, la responsabilité du maire, pourrait-elle être engagée, l'engagement d'une commune à réaliser la mise en oeuvre dans le cas du schéma communal suffit-il à protéger les élus lors de la campagne sénatoriale cette problématique a été soulevée par une très grande majorité des élus, je vous remercie pour votre réponse madame la ministre. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, la défense extérieure contre l'incendie et placé vous l'avez rappelé sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargés d'un pouvoir de police administrative spéciale cette défense, elle a pour objet d'assurer en fonction des besoins résultant des risques à courir l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et secours par l'intermédiaire des différents points d'eau identifiés à cette fin, je le rappelle, parce que c'est cela qui permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir rapidement et efficacement et dans des conditions optimales de sécurité qui puisse être transparente et su notamment des élus et des maires, la réforme de la DSI, qui a été conduite en 2015 à instaurer une nouvelle approche novatrice, elle ne répond plus à une norme nationale mais relève effectivement du règlement départemental élaboré par le préfet, cette réglementation, elle répond à un double objectif : renforcer la concertation avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la difficile dans la définition pardon et l'application des mesures qui sont mieux adaptés, nous souhaitons à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque territoire la distance maximale qui sépare les points d'eau et les risques à couvrir et déterminée au regard des enjeux locaux en matière de protection et des techniques opérationnel des sapeurs-pompiers cette fixation des distances elle déterminée par l'analyse du risque et elle conditionne d'ailleurs, les délais de mise en oeuvre, nous avons parfaitement conscience que cette réglementation qui est nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut-être parfois dans certaines communes et notamment rurales ce règlement, il peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables avec les retours de terrain j'ai souvenir quand j'étais moi-même élu local faire partie de ces commissions sécurité incendie, nous savons à quel point les retours de terrain, notamment des élus locaux que vous évoquez sont absolument fondamentaux en ce qui concerne la coexistence des règles d'urbanisme et des règles de défis, comme vous l'avez aussi évoqué et d'ailleurs la juridiction administrative l'a confirmé, il s'agit de 2 régimes juridiques distincts, il ne ne sont pas souhaitable d'établir une automate une automaticité pardon entre la présence ou le projet d'une construction et la présence obligatoire d'enfant doit d'incendie à proximité, cette nécessité, elle est donc lié à l'analyse des risques que nous avons évoqués et pas seulement à l'existence de la construction, je crois que c'est important de de le rappeler. Maintenant pour répondent particulièrement votre souci de protection des élus que nous partageons quant à un éventuel engagement de leur responsabilité en la matière, je voudrais rappeler que la réforme de 2015, ensuite à la mise en place des schémas communaux ou intercommunaux qui permettent de développer cette analyse du risque d'identifier les priorités et de les planifier sur plusieurs années, et d'ailleurs cette optimisation du déploiement de la DSI et son financement, peut aussi être obtenus en transférant le domaine aux établissements publics de coopération intercommunale, ce qui est le choix qui a été fait dans plusieurs endroits, dans certains cas strictement encadrées par la réglementation nationale un financement par des tiers peut d'ailleurs être envisagée la DCA à reposer sur un équilibre entre les impératifs de sécurité des populations sa constante amélioration le couch Nancy insupportable, notamment pour les communes rurales, le tout étant appréciée à l'échelon local, et elle est déployée depuis 6 ans, après des expérimentations positive notamment dans les Deux-Sèvres et en Ille-et-Vilaine, et ce bien avant 2015 ans comme vous le suggérez, le ministère de l'Intérieur envisage voudrait conclure une évaluation pour cette année, je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur, il vous reste 25 secondes si vous souhaitez répondre. Je sais pas grand chose à rajouter, merci madame la ministre, je crois que c'est important le la dernière phrase que vous avez cité concernant l'évaluation de la réforme afin de tenir compte des difficultés rencontrées par tous, elle est, par tous les élus des communes rurales, merci. Merci, cher collègue lors du jour appelle la question orale de Monsieur Cyril pelle va au ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, votre ministère a récemment annoncé qu'un décret venant réformer l'activité des sapeurs-pompiers volontaires étaient en cours de préparation pour une publication durant l'année 2021, ce décret aurait pour objectif de rendent le modèle français conforme au droit européen, notamment à la directive européenne sur le temps de travail et à prendre en compte l'arrêt massacre de la Cour de justice de l'Union européenne qui assimile les sapeurs-pompiers volontaires et des salariés, toutefois, cette réforme de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires viendrait totalement bouleverser le modèle français de la sécurité civile qui est basé sur l'engagement et le volontariat, elle aurait pour conséquence de soumettre les sapeurs-pompiers volontaires à des limitations en terme de cumul de temps de travail et empêcherait l'engagement de ces derniers, on sait qu'elle ne permettrait pas de dépasser 48 heures de travail hebdomadaire, temps passé entre astreintes comprises, cela viendrait donc limiter considérablement le nombre de personnes pouvant s'engager ferait passer le nombre de volontaires de 195000 à 48000 cette baisse drastique du nombre de pompiers viendrait faire peser un risque accru sur les administrés, tout particulièrement en période de crise exceptionnelle, tels que la crise sanitaire que nous connaissons actuellement par ailleurs la mise en oeuvre et de cette politique européenne viendrait obliger à embaucher des sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, ce qui représenterait un coût estimé à 2 5 milliards d'euros, les finances publiques étant déjà extrêmement mise à mal par des années de mauvaise gestion et par la crise sanitaire, il serait plus que malvenu que la France ait à supporter ces dépenses supplémentaires, en outre, le gouvernement s'est engagé à travailler sur l'élaboration d'une nouvelle directive européenne qui permettrait de protéger le volontariat, en matière de sécurité civile, solution qui sera bien plus adapté à la situation française que ce décret aussi, madame la ministre, pouvez-vous m'indiquer pourquoi votre ministère a commencé la préparation de ce décret, alors même que le gouvernement s'était engagé à ne pas le faire et à privilégier les négociations au niveau européen, avez-vous engager ces négociations et c'était le cas, quels sont les avancements allant dans le sens d'une nouvelle directive relative aux sapeurs-pompiers volontaires, qui ne bouscule qui ne bouleverserait pas le modèle français, vous engagez-vous à ne pas remettre en cause le fonctionnement français de la sécurité civile, on ne le faisant pas basculer vers un modèle basé sur le salariat des sapeurs-pompiers et enfin concernant le décret, pouvez-vous nous donner plus d'informations, le maximum de 800 heures est-il toujours d'actualité, est ce que les événements exceptionnels comme les feux de forêt seront prises en compte, seront comptabilisés, est ce que les astreintes seront-elles comptabilisées une heure pour une heure, autant de questions, Madame la Ministre, qui attendent vos réponses merci. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté pour 2 minutes 30. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, beaucoup de questions dans votre question, je pense que je ne pourrais pas répondre à tous dans le temps, qui met en partie mais je vous propose pas de poursuite des échanges ensuite si vous souhaitez à davantage de précisions, je voudrais vous répondre qu'il existe aujourd'hui un consensus partagé par une très grande majorité des acteurs sur la nécessité de pouvoir adapter ce modèle actuel de volontariat, non pas pour remettre en cause l'intégralité de son fonctionnement, alors qu'il a largement fait ses preuves, vous l'avez très bien rappelé tend au quotidien que dans les crises, mais au contraire pour travailler sur ce modèle que nous défendons collectivement à ce stade, il est utile de rappeler la position de la Commission européenne, qui a confirmé qu'elle n'envisageait pas de faire évoluer la directive 2003 88, celle du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ni de proposer d'ailleurs une nouvelle directive consacrée aux volontaires dans les services de sécurité civile, excluant de fait toute possibilité d'exclure formellement les sapeurs-pompiers volontaires du Champ de la déroute était telle qu'il a été envisagé avant par certains parlementaires, notamment donc c'est bien pour répondre à ce besoin de consolider notre modèle de volontariat, que le ministère de l'Intérieur a récemment initié des travaux de concertation qui doit faire naître suite aux échanges avec la Commission européenne de tirer les conséquences des problématiques qui ont été soulevées par certaines situations et de limiter, dès lors, les possibilités de qualification sapeur-pompier volontaire comme travailleur au sens de l'ADE tt, donc nous sommes vraiment loin d'une quelconque transposition aux sapeurs-pompiers volontaires de cette directive, ce que nous sommes convaincus qu'une fois ces ajustement réalisé le volontariat se trouvera de fait exclus du Champ de l'application de la de donc soyez assuré et rassuré, Monsieur le Sénateur, que les impacts que vous évoquez ne constitue en rien les éléments de la concertation qui débute la réflexion qui s'engage doit au contraire permettre d'avancer en liaison étroite avec les services d'incendie et de secours, et avec l'ensemble des acteurs partenaires et des élus pour disposer de leurs analyses sur ces problèmes, de leurs propositions en la matière, et d'ailleurs pourquoi pas également de vos propositions, mesdames et messieurs les sénateurs, parce qu'elles permettront d'alimenter par la suite, les travaux de consolidation de la réglementation voilà pour ce qui concerne ma réponse générale et comme je vous disais monsieur le sénateur, nous sommes à votre disposition vous répond, plus particulièrement, point par point à la suite de vos questions finales, je vous remercie.

Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Olivier Paccaud au ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame le Ministre depuis de nombreuses années, la sécurité routière est devenue une cause nationale et même si le bilan annuel reste toujours dramatiquement élevé avec plus de 3000 morts, nous sommes désormais bien loin des hécatombes des années 70 lorsque plus de 16000 de nos compatriotes perdait la vie sur les routes, tous les ans nos voitures sont devenus plus sur les routes sont aussi plus Secure la ceinture de sécurité, le permis à points, les limitations de vitesse, les campagnes de prévention, la pédagogie ont porté leurs fruits, la sanction aussi probablement par l'installation de radars cependant depuis quelques années un plancher semble atteint et le nombre de décès liés à la circulation ne baisse plus, par ailleurs, la multiplication des radars ne fait pas consensus et n'est plus ressentie par les Français uniquement comme un instrument de sécurité routière plutôt comme une arme fiscale déguisée, c'est ainsi que les radars sont devenus la cible prioritaire des gilets jaunes, voici 2 ans aussi alors que de nouveaux radars dits tours, elles sont en cours d'installation ne serait-il pas judicieux d'orienter une part minime 10 % par exemple des crédits consacrés à ces équipements vers la mise en place de radars pédagogiques bien moins coûteux mais tout aussi utile, certes ils ne rapportent pas un centime à l'État, mais il faut ralentir la plupart des automobilistes raisonnables n'est-ce pas là le but quand on sait qu'un radar pédagogique coûte en moyenne 2000 euros alors que la plantation radar retour elle est de plus de 32000 euros quand on sait aussi que de nombreux élus de petites communes souhaite sécuriser la traversée de leur commune via ces machines ne pourrait-on pas envisager la création d'enveloppes départementales via les préfectures spécifiquement dédiée à ces outils ne serait-ce pas là un bon moyen de démontrer à nos concitoyens que le gouvernement s'intéresse plus à leur sécurité qu'à leur portefeuille. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, les radars routiers sont d'abord un instrument de prévention, vous l'avez rappelé et d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre question, le but de ces radars, c'est justement de faire de la prévention, de faire ralentir et d'éviter un certain nombre d'accidents et donc la quasi-totalité des dispositifs de contrôle installés sont signalées par des panneaux très visible et les radars déployés dont le nombre a été limité à 4700 par une décision du comité interministériel de sécurité routière de 2015, d'abord une vocation préventive et j'insiste là-dessus depuis l'installation d'un 1er radar automatique en octobre 2003 le nombre des morts est passé de 5731 au cours de cette même année, à 3244 ans en 2019 en France métropolitaine, c'est sur quelques années, une baisse de 43 % une partie très significative de cette baisse et d'après les experts directement attribuée à la politique de déploiement de ces radars, donc s'il est vrai que ces radars ont aussi pour objet de permettre à la constatation des infractions aux règles de vitesse et la verbalisation de leurs auteurs, il constitue un élément fondamental de la politique de prévention des accidents sur la route, il est par ailleurs à débattre d'évoquer une multiplication des radars, si l'on regarde le nombre du déploiement de ceci, il y a eu, c'est vrai, un certain nombre de radars à remplacer, vous l'avez rappelé et à moderniser, entre 2000 19 et 2020, mais le programme des radars du Tour, elle en cours de déploiement n'a pas pour objet d'en augmenter le nombre, il en va de même pour le programme d'externalisation de la conduite de voiture radar déployés dans 4 régions : déploiement qui va se poursuivre en 2021 dans quatre nouvelles régions avec là aussi une vocation préventive ou de remplacement, enfin vous m'interrogez, Monsieur le Sénateur, sur les intentions du gouvernement concernant le comportement des conducteurs, je vous confirme que c'est bien notre intention d'inciter les usagers de la route, au-delà d'ailleurs des seuls conducteurs d'automobiles à adopter une conduite plus apaisée à partager plus harmonieusement, l'espace public et c'est cet esprit d'ailleurs qui inspire à la dernière campagne de communication de la sécurité routière, qui a été largement diffusé en télévision et sur les réseaux sociaux, qui rappelle que la transgression au quotidien des règles de sécurité routière se traduisent parfois par des drames et par des morts et c'est cet esprit qui guide quotidiennement les services de l'État, seule ou en concertation avec leurs partenaires notamment associatifs et élus locaux pour concevoir encadré organisé chaque jour sur le terrain, les actions d'éducation et de prévention sur les risques routiers dans les écoles, les collèges, les entreprises, permettez-moi de saluer leur engagement et leur mobilisation et de vous assurer monsieur le sénateur, que le gouvernement a fait ce choix de poursuivre cette politique de prévention et d'éducation routière : les radars n'en sont qu'une toute petite partie je vous remercie. Merci madame la ministre, monsieur le sénateur, il vous reste 35 secondes pour répliquer. Oui, madame la présidente, merci madame la j'ai bien entendu votre réponse, j'ai pas entendu parler des radars pédagogiques et je pense sincèrement qu'en matière de prévention, ils ont un rôle à jouer et la petite proposition modeste que je vous fais me semble mériter d'être examinés, parce que je pense sincèrement qu'il faut vraiment allié prévention et sanction efficacité et sagesse et faire confiance accorder un peu de responsabilité aux Français parce que très sincèrement et je le fais sans aucun cynisme sans aucune provocation, mais nos compatriotes pour eux radar ça rime avec piège avait pompe à fric avec tirelire et vous avez indiqué que les radars été indiqué. Pour les radars en tout cas dans mon département, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, et donc voilà peut-être aussi qu'il faut réhabiliter cette règle qui permet effectivement en entrée d'agglomération à certains automobilistes de ralentir. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Sylvie Vermeillet au 1er ministre. Merci madame la présidente, madame la ministre, j'attire votre attention sur le devenir des associations, la société des membres de la Légion d'honneur et l'association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite, suite à la diminution du nombre d'attribution des distinctions et la modification des critères d'attribution à l'issue du conseil des ministres du 2 novembre 2017, le 1er ministre a présenté une communication relative aux ordres nationaux par laquelle il a exprimé la volonté du président de la République d'engager une double révision de l'attribution des plus hautes distinctions nationales qui donne lieu à une réduction des effectifs, y a un respect plus strict des critères d'attribution et de leurs valeurs fondamentales, l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur récompense depuis leurs origines, les militaires comme les civils qui ont rendu des services éminents à la nation, pour la période 2018, 2020 le nombre de décorés est ainsi réduit pour la Légion d'honneur 5 mois 50 % pour les décors civils, moins 10 % pour les décorer militaires et moins 25 % pour les étrangers pour l'Ordre du mérite, moins 25 % pour les décorer civils, moins 10 % pour les militaires, et moins 20 % pour les étrangers, ces diminutions ne sont pas sans incidence sur les effectifs des 100 30 sections départementales de la société des membres de la Légion d'honneur et les 140 sections de l'association nationale des membres de l'Ordre national du Mérite, combiné au fait que de nombreux récipiendaires de la Légion d'honneur et de l'ONM n'adhère pas à leur association respective et au fait que celles-ci sont fortement touché par les décès de leurs adhérents vieillissant, les restrictions risquent d'accélérer l'érosion régulière constatée des effectifs des adhérents, ces associations, ces associations sont essentiels dans leur symbolique dans leurs actions de renforcement du lien intergénérationnel, elles disent-ils au quotidien les valeurs de citoyenneté et la transmission de la mémoire, je vous remercie, Madame la Ministre, de bien vouloir m'indiquer si une solution peut être apportée à ces associations menacées, sans quoi beaucoup d'entre elles pourraient disparaître à moyen terme. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, je vous réponds au nom du 1er ministre qui vous remercie pour votre question qui est l'occasion pour nous de rappeler notre attachement et notre respect pour nos 2 ordres nationaux la Légion d'honneur d'une part et le mérite, d'autre part, et c'est pour préserver leur prestige et leur qualité, que le président de la République grand-mère remettre de ces 2 ordres, a souhaité, dès son élection, engager une double révision des modalités de leur attribution par une réduction des effectifs, ce que vous avez rappelé mais aussi par un respect plus strict des critères d'attribution et des valeurs fondamentales de 16 hommes nous interroger sur les conséquences de ces nouvelles règles sur la pérennité des associations qui réunissent les récipiendaires de ses Oeuvres à la Société des membres de la Légion d'honneur et l'association des membres de l'Ordre national du Mérite, lesquels et je tiens à le souligner, même d'importantes actions au service de l'intérêt général, le gouvernement souhaite en 1er lieu souligner que ces associations sont parfaitement indépendante et que ni le grand maître ni le grand chancelier n'ont à connaître ni leurs actions, leur compte leur les ressources de ces associations proviennent d'ailleurs avant tout des cotisations des adhérents de d'Yverdon et legs et il aurait également loisible de faire appel à la générosité publique en sollicitant une subvention de l'État ou des collectivités territoriales, selon les procédures en vigueur, en second lieu, il nous semble important de rappeler que la baisse régulière des effectifs de ces associations, là je revendique par exemple 45000 membres contre les 55000 au début des années 2010, elle s'inscrit certes dans un contexte de diminution du nombre de récipiendaires mais surtout dans celui du vieillissement naturel des adhérents existants et d'un affaiblissement du taux d'adhésion à ces associations des nouveaux médias donc il conviendrait, à notre sens, de nous interroger en priorité sur l'attractivité de ces 2 associations pour les nouveaux médaillés sur les moyens de le renforcer à court terme, mais à moyen terme, comme par exemple, a commencé à le faire, la SML H avec son projet associatif, horizon 2030, qui met l'accent sur les activités à destination des plus fragiles et des plus jeunes, comme vous le savez, le gouvernement est confiant dans la capacité de ces associations à pouvoir faire face à ces évolutions, qu'il s'agit d'évolution réglementaire ou sociologique, elles ont montré par le passé, y compris d'ailleurs à la suite de réformes beaucoup plus drastiques des critères d'attribution comme lorsque le général de Gaulle avait décidé de plafonner le nombre de médaillés de la Légion d'honneur à 125000 alors qu'ils étaient au nombre de 320000 en 1962 et c'est un travail dans lequel évidemment le gouvernement, les parlementaires accompagneront ces associations, je vous remercie. Merci madame la ministre, chers collègues, vous avez 10 secondes si vous souhaitez répliquer. Merci madame la ministre, je crois que, eu égard au au respect que vous témoignez à à ces associations et à l'admiration que nous-mêmes nous nous leur porte. Moi, je suis plus inquiète sur le le l'évolution de leurs effectifs, et je ne saurais que vous vous recommander de d'examiner au cas par cas, association, par association d'évolution des effectifs et à leur apporter un soutien qui soit vraiment tangible, parce que la faiblesse de leur de leur effectif devient vraiment crucial merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Françoise Férat à la ministre de la transition écologique. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi mettant fin à la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en France vient de fêter son 3ème anniversaire le 30 décembre votre majorité l'a décidé : la France ne produira plus de pétrole et de gaz naturel à partir de 2040, ce taux découle d'une application stricte des accords de Paris sur le climat, issue de la COP21 signé ou engagés à l'être, par 194 pays dont acte, Nicolas Hulot, l'a affirmé dans cet hémicycle avec vigueur et certitude la France inspirera d'autres pays dans le monde, a-t-elle été suivie dans cette interdiction d'exploitation et de recherche, la France a-t-elle une perspective réaliste pour un monde sans pétrole et son gaz à partir de 2040, à à titre d'exemple, la société Exxon Mobil vient de découvrir au Guyana, ses 17ème et 18ème forages de pétrole, une production a déjà été démarré au rythme de 120000 barils par jour et une perspective de 220000 dès 2020 de fait notre loi se cantonne aujourd'hui à la fin du Made in France 2 questions précises, monsieur le ministre, qui attendent, je pense, de réponse précise quels sont les pays qui ont imité la France 3 ans après les accords de Paris, pouvons nous pouvons-nous parler de la fin des hydrocarbures dans le monde, dans moins de 20 ans, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari Ministre délégué chargé des Transports. Bonjour, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous interrogez, Barbara Pompili, qui, ne pouvant être présente m'a chargée de vous répondre la loi hydrocarbure, vous l'avez dit, est une mise en cohérence du droit français, avec nos engagements climatiques pris dans l'accord de Paris mais la France en conformité avec l'objectif de lutte contre le changement climatique, puisque pour rester en dessous de la limite des 2 degrés, il faut laisser la quasi-totalité des énergies fossiles dans le sous-sol la loi prévoit l'interdiction de l'attribution de nouveaux permis de recherche d'énergies fossiles, qu'il s'agisse du gaz de pétrole, ce qui mettra un terme à la recherche de nouveaux gisements et limite le renouvellement des concessions d'exploitation existantes à 2040, la production française d'hydrocarbures représentent aujourd'hui moins de 1 % de la consommation française et cette production a été divisée par 10 en 40 ans comme les gisements actuellement exploités s'amenuisent. Ne plus délivrer de nouveaux permis d'exploration conduit de fait à une extinction progressive mais plus rapide de la production nationale résiduelle d'hydrocarbures de permis d'exploration en cours de validité était relativement stable de l'Ordre de 60 il a fortement chuté depuis la loi hydrocarbures et ne compte plus que 17 permis actuellement d'ici à 8 ans il n'y aura plus de permis d'exploration d'hydrocarbures en France pour répondre à votre question, le Danemark et actuellement le second pays de l'Union européenne à avoir programmé récemment la fin de l'exploration et l'exploitation de ces ressources en hydrocarbures, notamment en mer du Nord, à horizon 2050 la France étudie sous l'égide de son représentant l'ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique, avec d'autres États la possibilité de créer une agence internationale pour une sortie du pétrole et du gaz, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, chers collègues, il vous reste un peu plus d'une minute pour répliquer. Oui merci madame la présidente, 194 pays, monsieur le ministre, et j'entends bien ce que vous venez de me dire : mais vous voyez-vous l'argument selon lequel on interdit d'abord chez nous et les autres suivront ne ne tient pas, ça paraissait évident évidemment très hasardeux, nous allons donc continuer à consommer des hydrocarbures pendant longtemps certainement de la, de 2040, bien sûr, je le regrette, autant que vous, cependant ils seront produits en dehors de nos frontières, dans des conditions environnementales que nous ne tolérerons pas chez nous et avec un bilan carbone importante pour le transport, nous avons le même objectif, monsieur le ministre, nous serons d'accord s'il plus une seule goutte de pétrole n'est utilisé, je ne défends pas le pétrole, vous l'avez bien compris mais tout simplement l'économie française, je vous remercie. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Corinne Imbert à la ministre de la transition écologique. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question portera sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de moulins ou le 30 juin dernier le 1er ministre de l'époque, Édouard Philippe, à accélérer le processus de destruction des moulins à eau en autorisant par décret le passage d'un régime d'autorisation, un régime de déclaration concernant la démolition des barrages, des moules cette démarche serait censé favoriser la préservation de certaines espèces aquatiques et ainsi présenter des vertus en matière de biodiversité et de continuité écologique sur le long terme, ces moulins à eau pour beaucoup, vestige de l'époque médiévale possède un potentiel non négligeable en matière d'hydroélectricité de plus ces aménagements demandés pour leur maintien sont particulièrement onéreux pour les propriétaires, enfin les moulins ou ont un rôle prépondérant en matière d'irrigation des plans d'eau conviendrait alors de s'intéresser aux véritables raisons qui menacent notre faune aquatique et non de pénaliser les propriétaires de moulins à eau acteur séculaire de l'équilibre entre l'activité humaine et la préservation de l'environnement ainsi ce centre 10000 et 20000 soldats et barrages qui pourraient être concernées à terme par des destructions. Aussi Monsieur le ministe, j'aimerais savoir si le gouvernement entend revenir sur cette décision et entreprendre une concertation visant à déboucher sur une solution respectueuse de l'environnement, de nos traditions et de notre Patrimoine historique n'est-ce pas une nouvelle fois une 7 une sur-interprétation de la directive européenne, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous interroger Madame Barbara Pompili qui ne pouvant être présente m'a chargée de vous répondre, la restauration de la continuité écologique des cours d'eau nécessite de concilier plusieurs enjeux, vous l'avez dit, qui sont parfois contradictoires, le gouvernement a lancé en juin 2018, un plan d'action pour une mise en oeuvre apaisé après une large concertation de toutes les parties prenantes priorisation des ouvrages meilleure prise en compte des enjeux patrimoniaux et sportif concertation renforcée implication des collectivités locales, financement de nombreuses actions sont en cours de déploiement. Dans un contexte de réchauffement des eaux et d'état critique pour la biodiversité aquatique, cette politique reste une priorité affirmée par les assises de l'eau en 2019, avec l'objectif de restaurer 25000 kilomètres de cours d'eau d'ici à 2022, à l'échelon européen, c'est l'une des mesures phares de la Stratégie Biodiversité pour 2030, le décret du 30 juin 2020 auquel vous faites référence n'est pas un décret anti-Moulin, il permet de simplifier les procédures en cours, améliorant la qualité des cours d'eau et des écosystèmes dans la logique d'accélération attendue par nos concitoyens, tous les petits barrages dont les seuils du Moulin peuvent avoir un effet significatif sur la migration des poissons les sédiments et les écosystèmes d'eau douce, il n'y a donc aucune raison objective d'exclure les seuils des moulins, les obligations de réduction de leurs impacts il n'y a cependant pas d'incompatibilité de cette ambition avec la sauvegarde de notre Patrimoine local lié à l'eau, différentes possibilités de restauration de la continuité écologique existe et la concertation locale permet d'identifier d'identifier la meilleure solution, au cas par cas en prenant en compte les contraintes et les opportunités locales qu'il s'agisse de la valeur historique et touristique ou énergétiques ou des usages de loisir de l'ouvrage considéré s'agissant plus particulièrement de la petite hydroélectricité de soutien à cette filière, fait partie des objectifs de la politique énergétique et afin de réduire les impacts environnementaux, la programmation pluriannuelle de l'énergie affiche une priorité à l'équipement de série existant dans le respect de la restauration des milieux aquatiques, plutôt qu'à la création de nouveaux seuils je vous remercie. Merci monsieur le ministre, il vous reste, chers collègues, un peu plus d'une minute pour répondre. Merci madame la présidente, merci Monsieur le Ministre, pour votre pour votre réponse, vous l'avez dit vous-même, il y a effectivement sur cette question, plusieurs enjeux contradictoires concernant la la migration des des poissons, vous le savez à l'endroit où il y a des moules où on il y a pas toujours possibilité d'avoir un contournement de du du de la rivière pour permettre à la fois le le le maintien et la préservation du du barrage du Moulin et à la fois faciliter la migration des des poissons, vous savez je suis je suis plutôt en général favorable à à la simplification, je me pose toujours une question : c'est quoi l'essentiel, cette question d'ailleurs vont devoir la poser pour toutes les politiques publiques qui sont, qui sont décédés, c'est quoi l'essentiel mais c'est vrai que cette ce décret de simplification, c'est une décision politique évidemment qui va contribuer tout de même à détruire des paysages et et un Patrimoine séculaires et c'est quand même donner les pleins pouvoirs à l'Agence de l'eau qui pourra se passer d'une enquête publique qui pourra se passer d'une étude d'impact pour arroser ses ces barrages et c'est, c'est là où ça me dérange sur le sur le votre remarque de la concertation locale, évidemment, je la partage, je pense qu'en effet il y a différents acteurs locaux, qu'ils soient politiques et administratifs qui sont les plus à même à déterminer ce qui doit être détruit ce que doit être, concert et les aménagements qui sont réalisés, je vous remercie, Monsieur le ministre et on on y regarde à 2 prix en Charente-Maritime, merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de notre présidente Annick Billon à la ministre de la transition écologique. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, la rénovation énergétique des bâtiments est un des piliers de la relance verte envisagée par le gouvernement pour tenir les engagements de la loi du 8 novembre 2019 relatives à l'énergie et au climat diminuer l'impact carbone des bâtiments poursuivent l'amélioration de leurs performances énergétiques et en garantir la fraîcheur pendant les étés caniculaires figurent parmi les objectifs de la future réglementation R 20 20 voulue ambitieuse et exigeante, l'intention d'appliquer l'indicateur de d'analyse du cycle de vie dynamique au sein de cette réglementation, apparaît comme une évolution favorable pour de nouveaux matériaux, ainsi la construction bois et les isolants biosourcés aura voix au chapitre du grand chantier pour lutter contre les passoires thermiques cependant cette évolution réglementaire aura une incidence majeure sur le développement de la filière qui nécessitera des investissements industriels conséquent pour pouvoir répondre à l'offre de marché des en investissement semblables à ceux effectués en Vendée, il y a déjà plusieurs années par des acteurs comme la coopérative agricole Caval pour le chanvre ou encore igloo pour la ouate de cellulose ou encore Hoffmann pour le ciment décarbonnées aussi, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, préciser dans quelle mesure le bilan carbone favorable des matériaux biosourcés sera pris en compte dans la réglementation revint 20 et quel plan de relance envisagez-vous pour aider les entreprises de la filière végétale, essentiellement des PME à investir afin d'augmenter la capacité de production française, je vous remercie. Merci président la parole est à monsieur Jean Baptiste Djebbari pardon, ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous interroger Madame Barbara Pompili qui ne pouvant être présente m'a chargée de vous répondre un contentieux oppose depuis plus de 20 ans, 2 fabricants de matériaux isolants représentative des 2 technologies l'isolant mince et les Wallons épais les performances respectifs de leurs produits en situation réelle de sont en question certains médias qui s'en sont fait l'écho, on évoqué à tort à scandale de l'isole Kate ce sujet aura toutefois eu le mérite de mettre en avant la nécessité que les conditions de pose des isolants respecte certaines règles pour que leurs performances soient pérennes, c'est pourquoi le gouvernement a conditionner la délivrance des aides pour l'isolation à la pose d'un système global d'isolation comportant également des dispositifs de protection est renforcé les critères de qualification RGE des entreprises qui pose ces isolant, la ministre du Logement a par ailleurs demandé de disposer d'éléments objectifs pour mieux connaître le comportement de ces matériaux dans la durée et le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, il travaille, s'agissant de l'élaboration de la prochaine réglementation environnementale 2020, des bâtiments neufs et revend, elle permettra d'aller plus loin que les précédentes régulation réglementation thermique, le ministère du Logement est en charge de définir les exigences de la future réglementation avec l'appui des meilleurs experts du domaine au CSTB à l'Ademe, il y a aussi RMA ainsi que des bureaux d'études indépendant sélectionnés par appel d'offres, menées ces derniers mois ont été très transparentes, elles ont fait l'objet d'un contrôle par des professionnels choisis au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, qui réunit l'ensemble de la filière, l'ensemble des contributions réalisé dans ce cas et public accessible, vous pouvez donc être assuré du plein engagement du gouvernement pour que l'aéroport soit donc le fruit de ce processus indépendant transparent et fondé sur une expertise reconnue au service du confort thermique dans les bâtiments et de la transition écologique, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez 43 secondes pour répondre. Merci madame la présidente, merci Monsieur le Ministre, pour cette réponse, vous avez prononcé le mot isole guettent, que je ne m'étais pas permis de de prononcer, vous avez parlé d'indépendance, de transparence, c'est ce que souhaitent les acteurs de ce secteur compte tenu des études qui sont que nous connaissons et de l'expertise que nous avons, nous savons que ces matériaux biosourcés que le bois ont des performances exceptionnelles, elles ne sont pas remettre en question, il ne s'agit, bien entendu, dans ce à travers cette question de ne pas opposer le minéral au végétal, de nombreuses entreprises sont déjà lancés dans cette transition avec ces matériaux, il est urgent de les accompagner, de mieux les accompagner plus près, je vous ai cité tout à tout à l'heure, 2 entreprises il y en a bien d'autres, je pense également aux établissements Kunio qui sont au coeur de notre cours ici au Sénat, d'ailleurs, et également à bois boréal à quoi donc, elles sont nombreuses, elles attendent votre soutien merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Catherine Morin-Desailly au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des Transports. Merci madame la présidente j'attire en effet l'attention de Madame la Ministre, sur l'évolution du projet du contournement Est de Rouen par la liaison à 28 à 13 chaque jour 40000 véhicules, donc ça ne 1000 poids lourds et 800 camions nocturne transportant des matières dangereuses sature les axes routiers de l'agglomération rouennaise face à la dégradation des conditions de vie qu'entraîne pollution Anne Both féerique et sonore aux entraves à la libre-circulation des habitants des communes limitrophes et à la paralysie de l'activité économique, l'État et les collectivités territoriales, au rang desquels la région Normandie dont je suis élue, mais également la métropole rouennaise et le département de la Seine-Maritime ont conclu en 2017, un contrat de 800 86 millions d'euros d'investissement pour ce chantier au-delà de l'intérêt pour moi la métropole rouennaise et leur désenclavement le contournement Est est avant tout un projet structurant majeur pour la Normandie, en effet, on constate aujourd'hui que la traversée de ce territoire et le goulet d'étranglement de l'axe autoroutier nord-sud ouest européen qui relie Stockholm à Gibraltar, la création de cette liaison à 28 à 13 connectera enfin la métropole rouennaise et donc toute la Normandie au reste de l'Europe une réelle chance pour l'économie du territoire métropolitain et pour la région, en tant que partie prenante, Monsieur le Ministre, l'État a également identifié l'intérêt stratégique que revêt le projet de contournement Est de Rouen on y apportons un investissement de 245 millions d'euros, en effet, celui-ci s'inscrit en complémentarité d'ailleurs du plan de relance présenté par le gouvernement en faveur des mobilités durables du fret ferroviaire et fluvial via l'axe Seine et des infrastructures de transport, le 19 novembre 2020, le Conseil d'État a rejeté sans ambiguïté les 13 requêtes déposées de contre le projet, relevant notamment que les études d'impact environnemental avait été particulièrement respectée, tous les voyants sont désormais ouverts aussi je souhaiterais savoir si l'État réaffirme bien cette nécessaire ambition est de connaître les intentions pour aider à faire aboutir ce projet, rapidement, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari Ministre délégué chargé des 30. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice bon Desailly vous m'interrogez à propos du projet de contournement Est de Rouen qui consiste, vous l'avez dit, on a tracé 9 de 40 kilomètres afin de relier les autoroutes à 28 et A13 et ainsi décongestionner la métropole rouennaise, je connais bien ce projet, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'en entretenir très récemment avec monsieur le maire de Rouen, ce projet a fait l'objet de nombreuses concertations depuis 10 ans la DUP a été délivré le 14 novembre 2017 après un avis favorable du Conseil d'État, vous l'avez rappelé les collectivités, partie prenante, la métropole de Rouen, le département de la Seine-Maritime, la région Normandie avait quant à elle confirmé leur engagement financier en 2017 pour 50 % de la subvention d'équilibre l'État a également confirmé son engagement correspondant à l'autre moitié du financement dans le cadre de la loi dans notation des mobilités ce projet autoroutier a en effet été retenu parmi ceux à engager dans la décennie et l'État se tient ainsi prêt à lancer la procédure de concession d'ici à fin 2022

de replanter 4 Oeuvres pour un déraciné, en outre, une attention particulière au suivi des nuisances sonores a été intégré le projet madame la sénatrice ne se fera pas contre les collectivités locales, nous avons besoin d'y voir clair rapidement sur la position de chacune d'entre elles, c'est pourquoi le préfet à notre demande, a demandé aux 3 collectivités partenaires de délibérer pour confirmer ce choix dans les semaines à venir, nous attendons à ce jour, le retour, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, chers collègues, vous avez 38 secondes pour répliquer. Merci, Monsieur le Ministre, parce que vous avez été très clair, vous avez réaffirmé l'intérêt stratégique majeur de cette infrastructure routière et en même temps vous avez levé toute question s'agissant de l'impact environnemental, donc vraiment je vous en remercie, au moment où, en effet, les choses sont en train de se conclure, le préfet a en effet demandé aux collectivités de se positionner le département, la Seine-Maritime, la fait il y a 4 jours, le 14 janvier dernier la réaffirmé fortement la région, il fera le 15 février la métropole le 8 mai il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent que ce projet s'engage aussi dans ce qu'on appelle de la transition écologique puisque forcément il s'accompagnera de toute une réflexion bien sûr sur les modes alternatifs et les modes doux, c'est un ensemble qu'il faut voir sur ce projet extrêmement important pour lequel vraiment, nous sommes un point très très très stratégique et cruciale, merci monsieur le ministre d'avoir réaffirmé la nécessité de ce projet. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Laurent Somon, transmise à la ministre de la transition écologique. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaite aujourd'hui vous alerter vous interroger au sujet du soutien de l'État aux acteurs de la filière gaz vers le plan de relance économique France relance de faire de l'écologie, l'une des grandes priorités du quinquennat et nous ne pouvons que toutes et tous nous en réjouir en effet réduire l'empreinte carbone est indispensable, alors pourquoi, entendons-nous trop souvent dans nos territoires que les délais sont trop longs, que les aides se sont attendus dans mon département de la Somme, la SAS agri-bioénergie a démarré la construction d'une unité de matinée après obtention des permis de construire et des autorisations d'aussi parce CPE au mois de septembre, et nous on voit aujourd'hui que partiellement le bout, 5 mois après, en effet, cette entreprise a rencontré une difficulté majeure qui a mis en péril l'issue est la concrétisation du projet de près de 7 millions d'euros après avoir sollicité depuis quelques mois, GrDF afin de pouvoir obtenir le contrat de raccordement au réseau, la SAS étaient toujours en attente de celui-ci à l'aube de l'ouverture du chantier, on leur avait pourtant assuré que pour le 15 octobre il disposerait du contrat, celui-ci étant bien sûr gage de validation au déblocage des fonds bancaires nécessaires à la construction cependant qu'elle ne fut pas leur surprise quand ils ont appris quelques jours plus tard que les règles de gestion d'accès au réseau de gaz avait changé depuis quelques jours, malgré le droit à l'injection et que dès lors, toutes ces dispositions et obligations sont désormais régi par la Commission de régulation de l'énergie, il y a, enfin, semble-t-il, de délibéré de manière positive sur ce dossier, cette lenteur, cette lourdeur administrative a ainsi l'ASS agri-bio énergies en situation de ne pas pouvoir régler ses fournisseurs et les premiers travaux étant effectué pour l'Ordre de 600000 euros, cette situation n'est pas la seule dans la Somme, ni même en France, alors soyons attentifs dans car, dans ce contexte de grave crise sanitaire et économique, il paraît inconcevable de laisser les sociétés agricoles abandonner ses projets vertueux, d'autres attendent confirmation des subventions de l'Ademe, qui conditionne la finalisation du plan de financement de leurs projets, entre-temps, une autre annonce gouvernementale est venue perturber la filière en effet à la fin de l'année dernière Madame la ministre de la transition écologique déclaré qu'à l'été 2021, il ne sera plus possible de construire de nouvelles maisons individuelles exclusivement chauffés au gaz, comment donc expliquer à ceux qui investissent pour produire du gaz vers que les habitations neuves ne pourront plus, quant à elle être chauffé au gaz d'un côté nous incitant les Français à produire et consommer, d'une manière vertueuse alors que de l'autre, on va les empêcher de se chauffer au gaz, je ne suis aujourd'hui le porte-voix de toutes ces structures agricoles qui peine à voir le dossier avancer, j'ai le Ministre, vous le savez, beaucoup de nos concitoyens d'agriculteurs au rendez-ont des difficultés ne se relèveront pas ma question est donc simple : il il y a-t-il une réelle volonté à court terme, de développer les ENR issus de la biomasse et que comptez-vous faire pour aider ces entreprises et plus largement la filière agricole qui souffrent pour lesquels la méthanisation et source la diversification et pour les territoires, source d'autonomie énergétique et de production qui air d'énergie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur vous interrogez Madame Barbara Pompili qui ne pouvant être présente m'a chargée de vous répondre, le gouvernement est pleinement engagée dans le développement de la filière de production du biométhane créée en 2018 par la loi, agriculture et alimentation, le dispositif d'aide au renforcement des réseaux fait partie des dispositifs mis en 9 pour soutenir cette filière, ce dispositif permet de faciliter le raccordement des projets d'installations de production de biométhane à réseau gazier en faisant supporter les coûts des renforcements nécessaires des réseaux de gaz naturel par le biais des tarifs d'utilisation de ces réseaux plutôt qu'aux producteurs de biométhane l'objectif ambitieux de développement de la production de biométhane passe par un usage efficient et maîtrisée des dispositifs de soutien, il s'agit de la raison pour laquelle le dispositif d'aide au renforcement des réseaux comprend un mécanisme de vérification par la Commission de régulation de l'énergie, la crue de la pertinence des projets de renforcement, la Creuse, vous l'avez évoqué, a mis en place un mécanisme de vérification portant sur des zonages de raccordement ces zonages vise à rechercher pour chacun des territoires concernés le schéma de réseau le plus pertinent pour le raccordement des installations de production de biométhane si un délai est initialement nécessaires pour l'élaboration des zonages ces zonages permet ensuite de faciliter et d'accélérer la vérification des projets de renforcement des réseaux de gaz naturel nécessaire pour le raccordement d'installations de production de au cours des 6 derniers mois, ce sont d'ores et déjà 150 zonage qui ont été validés par la Commission de régulation de l'énergie, une nouvelle délibération étant prévues cette semaine pour une quarantaine de zonage additionnel, cela représente cumulativement un investissement d'environ 100 millions d'euros, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, l'ordre du jour appelle la question orale du sénateur Fabien Gay au Ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des Transports. Merci, merci, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Seine-Saint-Denis jouxte Paris et pourtant il s'agit d'un territoire dont certaines zones sont totalement enclavé, parce que l'offre de transports en commun étaient insuffisantes et couvre mal le territoire, vous le savez, Monsieur le Ministre, ainsi le RER B et nous parlons en connaissance de cause puisque beaucoup de nos collègues du groupe CRCE en leçon usagers quotidiens transporte près d'un 1000000 de voyageurs par jour, ce qui en fait la 2ème, ligne d'Europe, or cette saturation entraînent des incidents, des ralentissements et des retards à répétition et ces incidents ne sont pas sans conséquences pour les usagers, notamment dans leur vie professionnelle et personnelle ou les retards viennent lourdement les handicapés en conséquence de cette offre de transport insuffisante l'utilisation de véhicules personnels occasionne un engorgement des routes et notamment de l'autoroute A1, avec la pollution qui l'accompagne ainsi à titre d'exemple, 76 % des salariés de la zone aéroportuaire Charles-de-Gaulle utilisent leur véhicule pour les trajets du domicile au travail, l'amélioration de l'offre et de transport et donc fondamental pour le quotidien des ces quoi d'Niger c'est particulièrement le cas des Tremblaysiens les Tremblaysiens qui attendent la nouvelle ligne 17 du métro car cette ligne permettra de désengorger les transports existant, l'autoroute est de fournir une alternative aux salariés des bassins d'emploi du parc des expositions d'Aerolia et de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, certes, nous pensons qu'il faut abandonner la station du triangle de Gonesse, située en plein Champ, et dans une zone interdite à l'habitat, non seulement pour laisser ces Terres fertiles à des projets respectueux de l'environnement, mais également afin de ne pas ouvrir la voie à de grands projets de construction nocif pour l'environnement et nous pensons à Europa City, en revanche, la ligne 17 dans son ensemble et hormis cette station est absolument nécessaire, aussi Monsieur le Ministre, les Tremblaysiens Tremblaysiens mais également tous les territoires concernés par le parcours, la ligne 17 et ses correspondances ont besoin de savoir si le calendrier initial de mise en circulation de la ligne 17 pour 2030 est maintenue et si la mise en service de la station Parc des Expositions Tremblay-Villepinte est toujours prévue pour 2028 si ce calendrier n'était plus d'actualité, quelles sont les nouvelles échéances Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur gay vous interrogez le gouvernement à propos de la réalisation de la ligne 17 notamment, et du futur métro Grand Paris Express, ce projet est en effet une priorité du gouvernement et des acteurs locaux le Grand Paris Express est un projet qui avance voudrais préciser ici que plus de 40 kilomètres sur les 200 ont déjà été creusés et que 20 milliards d'euros sont engagés, à cet égard les premiers tronçons devraient être livrés entre 2024 et 2030 et je reviens dans un instant, sur ces sujets de de calendrier, la crise sanitaire que nous traversons, a évidemment impacter son échéancier de réalisation, nous travaillons notamment sur des scénarios alternatifs afin que le 1er tronçon de la ligne 16 entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget, RER, soit par exemple bien ouvert pour les Jeux olympiques de 2024, des études sont en cours afin de réévaluer les priorités et le phasage du projet, les résultats seront connus d'ici à l'été prochain, concernant la ligne 17 j'avais annoncé l'été dernier le report après les JO de son 1er tronçon entre Le Bourget, RER et Le Bourget, aéroport, par ailleurs, comme vous le savez, il convient de rester attentif aux suites d'un recours contentieux contre l'autorisation environnementale de la ligne 17 qui pourrait compromettre les échéances, ainsi, s'agissant des autres tronçons entre Le Bourget, aéroport et le Mesnil-Amelot, il est encore un peu tôt pour évaluer les impacts éventuels de la crise sanitaire et du contentieux en cours sur les échéances de mise en service prévue à ce jour, entre 2027 et 2030 selon les sections, vous l'avez rappelé toutefois je peux d'ores et déjà vous confirmer que la réalisation de la ligne 17 est maintenue telle qu'elle est prévue au schéma d'ensemble du Grand Paris, cette ligne de 27 kilomètres traversera bien les 13 communes dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne et facilitera le quotidien de près de 565000 habitants, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, vous avez. Une poignée de secondes pour répondre à 9 secondes 9. Je vais essayer de réaliser cet exercice seul ministre non, juste une question, je vous remercie pour votre réponse, mais ce qui n'est pas entendable c'est que vous nous dites, le Covid a ralenti les travaux malheureusement il a pas Roland Petit, le Charles-de-Gaulle Express parce qu'en pleine crise du Covid vous avez relancé les travaux du Charles-de-Gaulle Express il faut abandonner cette ligne mettent les moyens pour les usagers du RER B et finir toutes les lignes du Grand Paris, parce que les habitantes et les habitants de la Seine-Saint-Denis ont droit à l'égalité républicaine, et à des transports en commun de qualité, ils payent leur passe Navigo au même type que les Parisiens au même tarif et ils ont droit à une hausse de transport de qualité comme les autres, je vous remercie. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Pierre-Jean Vergnes ELN au Ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des Transports. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la virgule Roissy la virgule, Roissy c'est un projet d'un tronçon ferroviaire de 6 qui permettra de raccrocher Roissy à la ligne de chemin de fer Paris-Soissons, Laon, Hirson. L'intérêt, il est pour les Axonais de pouvoir avoir accès à Roissy et à ses zones d'activité, donc d'y trouver d'y trouver du travail, l'intérêt, il est pour ceux qui arriveront à Roissy et qui pourront, dans le temps, utiliser cette ligne pour aller visiter la nouvelle Cité internationale de la francophonie, ce projet ses 6 kilomètres, c'est un enjeu structurant, essentiel et vital pour le sud de l'haine et pour l'ensemble du département de laine, on sait qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de dossiers lourds qui ne font pas toujours l'unanimité, là on peut dire, pour le coup que les élus et tous les acteurs sont derrière ce projet dans le CPER actuels, il y a une somme de 150000 euros qui est fléchée pour la réalisation des études participe, la région et auquel participe l'État ma question Monsieur le Ministre, c'est de savoir si vous pouvez, réaffirmé la volonté du gouvernement d'inscrire dans le prochains CPER les travaux de raccordement et de 7 Roissy et tant que je suis sur les CPER savoir le délai dans lequel les CPR seront signés entre les départs entre les régions et l'État, merci de vos réponses. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean Baptiste Djebbari Ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vert je veux vous assurer de mon attention toute particulière au désenclavement des territoires peu desservi par les différents modes de transport pour connaître bien le sujet, les transports du quotidien sont au coeur de la politique de ce quinquennat et le mode ferroviaire fait l'objet d'un soutien sans précédent j'ai bien pris acte du souhait des élus locaux, d'améliorer la desserte ferroviaire entre l'est et l'Île-de-France, toutefois, la question d'un nouveau barreau ferroviaire entre la ligne Paris-Laon et la ligne à grande vitesse d'interconnexion menant à l'aéroport Roissy- Charles-de-Gaulle se pose à plus long terme, l'opportunité de ce projet a été analysée dans le cadre d'une étude exploratoire sur l'accessibilité de l'aide à l'Île-de-France, menée en 2013, dans le cadre du CPE, vers 2007, cette dernière avait notamment évoqué plusieurs pistes d'action dont la réalisation de ce nouveau barreau pour un coût minimum de 110 millions d'euros, mais aussi l'amélioration des dessertes et des correspondances avec le réseau francilien, ou encore celle de l'infrastructure de la ligne Paris-Laon dans la continuité de cette première étude, j'entends la nécessité de mettre à jour et d'approfondir l'analyse fonctionnelle et technique d'Intel à à ce titre, je vous confirme l'engagement de l'État, aux côtés de la région de France à hauteur de 150000 euros en 2021 pour financer l'étude correspondantes ce financement démontre l'attention que l'État porte, développement économique et à l'attractivité du territoire axonais cette étude viendra également alimenter les réflexions globales à conduire pour l'ensemble des opérations prévues sur le réseau Nord en particulier au sein de la plateforme, services et infrastructures dédiées réunissant toutes les parties prenantes, État, collectivités et SNCF, réseau sur cette partie du réseau, comme vous le savez, le président de la République et le gouvernement ont d'ores et déjà définis comme prioritaires pour les 5 années à venir, le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie dont l'enquête publique se tiendra au 1er trimestre 2021, je vous remercie. Merci monsieur le ministre, chers collègues, il vous reste une minute pour répondre, si vous le souhaitez. Merci, nous passons donc cas à la suite de l'ordre du jour qui appelle la question orale de Monsieur François Bonhomme, transmise à la ministre de la transition écologique. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, ma question porte sur le projet de territoire du bassin versant du desk ou à un particulier de la rotule, le projet de retenue de Sylvain sur ce site a été abandonné en catimini en 2015 depuis les institutions écologiste, les agriculteurs des syndicats agricoles, les élus et membres de l'instance de dite de co-construction tentent de trouver un consensus sur ce dossier devenu sensible les 4 ans qui viennent de s'écouler près de 200 réunions et groupes de travail se sont succédé et pourtant la décision tarde toujours à venir, chacun s'accorde cependant reconnaître existence de tensions sur l'eau et les milieux aquatiques le territoire et les cours d'eau qui sont, en effet, en souffrance depuis de nombreuses années, à l'image de la qualité de l'eau du desk ou médiocre en qualité et en quantité, il est donc indispensable de trouver les moyens d'une gestion équilibrée de la ressource à nous sur ce secteur, 5 ans après le projet demeure au point mort alors qu'il se relève, révèle de plus en plus nécessaire pour clarifier les besoins agricoles des départements de Tarn-et-Garonne et de Tarn qui représenterait plusieurs dizaines d'agriculteurs d'agriculteurs ce ce territoire, je vous demande donc de bien vouloir me dire : Monsieur le Ministre, les mesures envisagées par le gouvernement pour lancer enfin une phase opérationnelle, c'est-à-dire une phase de réalisation pour permettre une meilleure gestion des ressources sur ce secteur. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean Baptiste Djebbari Ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur vous interrogez Madame Barbara Pompili qui ne pouvant être présente m'a chargée de vous répondre, je tiens tout d'abord à saluer le travail de concertation mené ces dernières années par l'ensemble des parties prenantes ayant permis après la mort tragique de Rémi Fraisse, donner un un sens à l'après Sivens à travers un nouveau projet de territoire pour la gestion de l'eau sur le bassin versant du Tesco, le projet initial avait provoqué de vives contestations locales car elle prévoyait de stocker 1,5 millions de mètres cubes d'eau pour de l'irrigation et du soutien d'étiage et aurait conduit à la destruction de 13,4 hectares de zones humides dans cette configuration initiale, il a été abandonné par le conseil départemental qui a été indemnisés par l'État, un nouveau cadre de réflexion préalable à la construction d'un ouvrage a donc été défini basée sur la concertation locale, alors où en sommes-nous aujourd'hui conformément au processus de concertation promise par le gouvernement, les travaux menés ont permis d'établir un diagnostic de la ressource en eau disponible, de préciser les besoins pour l'agriculture en s'inscrivant dans une logique de transition agro-écologique de recherche de valeur ajoutée de revenus satisfaisant pour ce territoire majoritairement de petites exploitations en cultures élevage avec des revenus modestes, comme le démontrent les différentes études, il reste aujourd'hui à finaliser les discussions sous l'égide de la préfète et de l'Agence de l'eau, la ministre a entendu l'impatience de certains acteurs et nous la comprenons mais la concertation qui s'est tenu ces derniers mois, mérite de prendre le temps d'aboutir sur un compromis à la hauteur du travail accompli la ministre tient à réaffirmer son engagement et celui du ministre de l'Agriculture quant à la mise en oeuvre opérationnelle d'un nouveau projet de territoire conciliant enjeux environnementaux et agricoles, s'agissant de la création d'un ou plusieurs ouvrages pour mobiliser la ressource en eau, en complément de l'optimisation des retenues déjà existantes et d'économie d'eau, le volume d'eau stockée devra être calibré au plus juste en réduisant ses impacts sur le milieu, ce que la loi permet je vous remercie. merci Monsieur le Ministre, l'historique vient d'être faite, ce n'est pas simplement le comité départemental qui annulé, c'est l'État en catimini qu'a pris un arrêté d'abandon et tenez-vous bien, le 24 décembre 2015 ne trompe pas : on arrêté le 24 décembre c'est qu'on ne cherche pas beaucoup à faire de la publicité d'une part depuis, depuis il ne s'est pas passé grand chose alors on a été consensuel, on a fait une instance dite de co-construction selon la mode actuelle on a représenté, on a reconnu des groupes écologistes de la représentativité, être vraiment un sujet à caution et depuis on a fait 700000 euros d'études supplémentaires alors que les études préalables avaient déjà été faites les les instincts de construction présidée par 2 élus ont fait des propositions consensuelles qui ont été mis sur la table et depuis on attend toujours que l'État tranche il ne tranche pas bien sa responsabilité, je rappelle que l'enjeu, c'est quand même l'irrigation si de permettent de logements de territoire et le temps que nous perdons à cela est très préjudiciable, monsieur le ministre, au aux agriculteurs qui attendent et qui se fatigue qui se fatiguent et ne faudrait pas joué une espèce de de jeu théâtral ou dans lequel, à force d'épuisement, on finit par tout renoncé. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Christine Bonfanti Dossat au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame le la présidente, monsieur le ministre je suis interpellé par le SAMU d'un suite à de récentes décisions de l'ARS de Nouvelle Aquitaine qui a décidé de restreindre la collaboration des médecins libéraux aux soins du centre de réception et régulation des appels du SAMU se seulement aux interventions COVID 19, monsieur le ministre, lorsqu'un système fait ses preuves, le bon sens commande de lui octroyer les moyens humains nécessaires pour se renforcer en temps normal comme en temps de crise, la collaboration exemplaire ville hôpital au sein de ce centre de régulation a fait ses preuves, pourtant aujourd'hui elle est mise à mal les personnels du SAMU 47 de comprennent pas les récentes décisions de l'ARS et je ne me joindre à leur incompréhension, faut-il vous rappeler que les bêtes saines urgentistes sont déjà soumis à une activité à flux tendu, non seulement au SAMU mais dans leur exercice au quotidien aux urgences de l'hôpital d'Agen et pour le SMUR d'gène et de Nérac, l'intervention de leurs collègues généraliste est donc primordial. La possibilité de voir retirer des plages horaires en régulation médicale pour la médecine libérale deviendrait alors un véritable non-sens en laissant ses décisions perdurer, c'est en même temps l'expertise, l'expérience, le savoir et les passions que vous tuer à petit feu le SAMU du Lot-et-Garonne est un modèle de réussite seul SAMU de France qui gère de façon autonome et partagée, l'articulation territoriale toutes les nuits et, parfois, et parfois la journée en assurant aussi la régulation supra-départementale pour le Gers en lieu et place des médecins du SAMU 32, alors Monsieur le Ministre, même si nous savons que cette organisation sera pérenne, jusqu'au 9 février puisqu'elles viennent d'être rallongé quelle décision comptez-vous prendre pour donner à ce centre de régulation, les moyens humains nécessaires à son bon fonctionnement. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Madame la présidente, madame la sénatrice Christine Bonfanti Dossat avant de vous réponde sur votre question, alors qu'un mouvement de libération de la parole important à court sur les réseaux sociaux avec tout inceste permettent de rappeler le déplacement que j'ai fait à agent dans la maison du Docteur Jean Bru qui la seule structure en France qui s'occupe de jeunes filles victimes d'inceste poignant des échanges que j'ai pu avoir avec certaines de ses pensionnaires, plus précisément sur la question que vous évoquez, s'agissant du SAMU, vous le savez, les difficultés des structures d'urgence sont pour partie. Il y a l'augmentation continue du monde de passage qui a doublé en 20 ans dans le dans le territoire mais aussi à la démographie des médecins urgentistes et aux difficultés de trouver, dit des lignes nous y répondons par le déploiement du pacte de refondation des urgences. Qui était réaffirmée dans le Ségur de la santé récemment et de ses 12 mesures clés, je pense notamment à la question de la coordination entre hôpital et médecine de ville, vous savez que c'est un des enjeux clé qui fait ses preuves depuis le début de la crise sanitaire je je le crois en ce qui concerne votre territoire, plus précisément, des mesures de soutien ont été apportées au SAMU centre 15 par l'Agence Régionale de Santé dès le début de la crise en février, l'ARS validait un renforcement de la régulation libérale notamment étendu à des périodes hors horaires de permanence de soins ambulatoires et avec un forfait de régulation qui a été revalorisé sur cette tranche horaire qui est passé de 70 à 92 euros de l'heure, ce dispositif exceptionnel a été prolongée jusqu'à ce jour dans la mobilisation des médecins libéraux s'est avérée précieuse pour faire face à l'augmentation du nombre ces mesures de soutien sont traduites par un effort financier majeur à hauteur de 2 millions d'euros sur la période de mars à décembre 2020 en région nouvelle Aquitaine, soit une augmentation de 25 % de l'enveloppe régionale qui est dédié à la régulation libérale en temps normal, dans le Lot-et-Garonne, cela représente une hausse de 46 des moyens qui sont consacrés chaque année fin de pouvoir adapter les ressources, on regarde l'évolution de la situation, l'ARS a mis en place un dispositif dédié de suivi de l'activité des SAMU centre 15 en lien avec l'Observatoire régional des urgences des indicateurs de suivi, ont été mises en oeuvre, reposant sur des données qui sont remontées quotidiennement par les SAMU des pics d'appels ont bien sûr été identifiés mais sur la période septembre décembre l'activité globale de régulation a plutôt diminué par rapport à l'année précédente, au niveau du SAMU 47 par exemple, l'activité et ainsi de 15 % inférieure à celle constatée en en 2019 toutefois, compte tenu des incertitudes importantes qui concerne l'évolution de la situation épidémique et du risque de rebond, l'ARS a décidé de maintenir les renforts de régulation a loué jusqu'à présent, une réunion de concertation est prévue le 9 février prochain qui permettra de partager ce diagnostic sur la bonne adaptation des moyens : l'évolution de la crise sanitaire voilà madame la sénatrice pour ces éléments de réponse. Il monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il vous reste 26 secondes. Merci, Monsieur le Ministre, d'abord de vos propos encourageants concernant votre visite et merci encore d'avoir fait le déplacement, alors je vous venez de répondre en disant qu'effectivement jusqu'au 9 février il y aurait donc une clause de revoyure pour prendre une décision, moi, je crois, monsieur le ministre, qu'il faut tuer dans cet hémicycle, la modernité à tout prix, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui fonctionne bien et donc, par conséquent, je serai très attentive au delà du 9 février de de savoir et devenir un soutien total avec le personnel du SAMU 47 qui bien sûr souhaiteraient vivement que cette organisation se poursuivent. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de la présidente Laurence Rossignol au secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la Santé, chargée de l'enfance et des familles. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, vous avez le 28 septembre dernier prononcer un discours sur les 1000 premiers jours de l'enfant, plusieurs des mesures annoncées à cette occasion, été très bien accueillie par les professionnels de la petite enfance, notamment par les assistantes maternelles et je pense tout particulièrement aux 45 millions d'euros consacrés à un plan de formation pour les professionnels de la petite enfance et à l'annonce d'une amélioration à la fois de la rémunération et des conditions de travail des assistantes maternelles mais vous le savez la crise sanitaire a laissé des traces dans cette profession, en particulier le premier confinement qui a aggravé des sentiments de manque de reconnaissance, d'abandon d'indifférence à leur profession, elles ont fait face au début un manque d'informations à des difficultés pour accéder à du matériel pour protéger les enfants et se protéger ainsi que leurs familles, et puis il y a eu sur la question de de la hauteur de prise en charge du chômage partiel d'abord 80 au lieu des 84 % de droit commun, puis ensuite une annonce de 84 % pour les actions de maternelle, puis ensuite une année, cette annonce a été remise en cause et le sujet est toujours en cours de discussion, les difficultés des assistantes maternelles pendant la crise, on était grande aux sciences qui concerne leur situation financière difficultés droit, de droit au chômage, difficulté de rompre un contrat pour non-paiement des heures de travail ou pour le non plus non paiement également des sommes dues par les parents, alors, alors qu'il bénéficient de CMG calcul imprécis des abattements fiscaux, bref, vous connaissez le dossier, vous le portez, vous vous y intéressez vous voulez le faire avancer, comment comptez-vous poursuivre les discussions avec les assistantes maternelles sur la revalorisation et la stabilité de leurs revenus, et enfin une petite question subsidiaire, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si les personnes de la petite enfance, crèches et assistantes maternelles sont incluses dans la stratégie vaccinale du gouvernement et à quelle étape, ils seront concernés. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. des familles. Non, madame la sénatrice Laurence Rossignol. Je partage évidemment votre préoccupation vers les les assistants maternels qui ont été, vous l'avez rappelé durement éprouvée par la crise épidémique, notamment dans sa première phase dès ma prise de fonction a coïncidé avec la seconde phase, avec le second confinement, j'ai été en contact avec elle de façon régulière, comme avec l'ensemble des professionnels, protection de l'enfance également pour les accompagner au mieux et que ce soit d'ailleurs pour moi l'occasion de saluer à nouveau leur engagement et de redire mon attachement à l'accueil individuel, qui est une composante singulière et essentielle de l'offre française des modes d'accueil du du jeune enfant, alors je me réjouis de savoir que vous approuvez plusieurs des mesures effectivement qui ont été annoncées en faveur des assistants maternels que j'ai qui remonte à septembre dernier, vous l'avez rappelé depuis cette date, d'autres annonces sont venus et préciser ou les compléter, notamment à l'occasion du dévoilement des grands arbitrages pris dans le cadre de la réforme du cadre normatif applicable aux modes d'accueil du jeune enfant, je pense par exemple à l'ouverture aux assistants maternels du bénéfice de la médecine du travail revendiquée de longue date par les représentants de cette profession, et on peut légitimement comprendre pourquoi vous évoquez aussi les dispositions de l'article 100 de la loi d'accélération et de simplification de la loi de l'action publique, la loi dite ASAP

je souhaite en 1er lieu rappeler que cette plateforme rénovée permettra d'une part aux parents d'avoir une vision plus claire et plus fluide de l'offre d'accueil à leur disposition et, d'autre part aux assistants maternels de pouvoir pour certains accéder plus facilement à des parents employeurs, c'est donc une évolution qui, me semble-t-il, est au bénéfice de tout le monde, en second lieu, je tiens à vous rassurer concernant les inquiétudes qui est que vous avez résumé qui ont été soulevées à l'occasion du projet de loi de finances pour 2020, après consultation des représentants de la profession, le texte qui a été proposé au Parlement avait été modifié par le gouvernement, sur 2 points. D'abord, et même s'il a été maintenu l'obligation pour les assistants maternels de s'inscrire sur ce site d'être communiquées aux gestionnaires du site leur adresse, il n'y aura pas d'obligation à ce que cette adresse soit publié l'instant maternelle pourra opter pour qu'une seule indication de distance au domicile des parents soient communiqués en ensuite le texte, voté, garantit que le fait de ne pas renseigner ses disponibilités ne constituera pas à soi seul un motif de retrait d'agrément, c'était une des grandes inquiétudes et là aussi je comprends pourquoi, voilà enfin et quant au manque d'ergonomie du site simplement vous dire que la Caisse nationale d'allocations familiales qui, éditrice du site a conscience que les services actuels ne donne pas satisfaction, un chantier de rénovation du site est actuellement menée avec des parents et aussi avec des assistants maternels volontaire et la CNAF s'adressera prochainement, a présenté ses évolutions associations pour terminer je termine mène à la présidente sur votre toute dernière question subsidiaire sur la place des des personnels de la petite enfance de la stratégie vaccinale, vous savez que notre stratégie est fondée notamment sur une priorisation progressive en fonction de l'Exposition des différents publics au virus et de leur sensibilité, d'où les personnes n'en est pas de d'où les personnels soignants en contact avec ces personnes et nos concitoyens de plus de 75 ans, comme la population générale, le moment viendra pour les personnels de la petite enfance, mais d'être vacciné et nous l'espérons, le plus tôt possible, le gouvernement en toute transparence, comme depuis le début, communiquera à cet égard. Secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Bernard Bonne au ministre des solidarités, de la santé. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, ma question concerne la nécessaire revalorisation des visites à domicile assurée par les médecins généralistes auprès des patients Covid. Nos hôpitaux ont fait face ces derniers mois, la violence de la reprise de l'épidémie Covid 19 et certains sont au bord de la rupture, notamment dans mon département de la Loire, nous craignons aujourd'hui une nouvelle flambée accentuée par la présence sur notre territoire de différents, variant face à cette arrivée massive et continue de malades, il faut impérativement désengorger nos services hospitaliers et notamment les services de réanimation. C'est pourquoi monsieur le ministre, il est urgent d'impliquer la médecine libérale, en particulier les médecins généralistes dans le suivi des patients Covid 19 qui sont stabilisés et ont quitté l'hôpital, que ce soit dans des structures spécialisées type iPad ou surtout à domicile dans le cas de la du Ségur de la santé, le ministre avait indiqué que les professions libérales devait négocier directement avec l'assurance maladie pour les revers déjà revalorisations tarifaires, or l'article 33 du PLFSS propose de reporter à 2023 les négociations conventionnelles, par ailleurs, la cotation qui prévaut pour les actes de visites à domicile, suite à un décret d'avril 2020 permet en Ephad de côté, à un niveau plus élevé ces visites, il y a là une véritable injustice pour la prise en charge des patients Covid 19 stabilisé, il paraîtrait tout à fait normal que les médecins généralistes, acceptant de prendre en charge le suivi à domicile de ces pathologies lourdes puissent eux aussi bénéficier de cette dérogation tarifaire ou de bénéficier d'une lettre-clé permettant une valorisation de ces actes de visites à domicile aussi Monsieur le Ministre : quelles mesures entendez-vous prendre pour accompagner les médecins généralistes qui accepterait, dans le contexte fortement dégradée sur le plan sanitaire que nous connaissons de prendre en charge les patients Covid au sortir de l'hôpital. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Bernard Bonne, vous m'interrogez sur la nécessité d'une revalorisation des visites à domicile auprès des patients atteints de la COVID 19 assurée par les médecins généralistes et une plus grande association de de ceux-ci à la politique mise en oeuvre, je pense pouvoir parler au nom et je sais pouvoir parler au nom du du ministre Olivier Véran vous disant que nous sommes évidemment très attentifs au remarque que vous formulez pleinement conscient du rôle fondamental de la médecine de ville, sur le même modèle que pour les interventions en n'est pas de professionnels de santé, des mesures dérogatoires ont été prises à destination des patients qui ne résident pas en établissement, il s'agit notamment de la prise en charge à domicile par des médecins de ville, des patients atteints de la COVID 19 ne nécessitant pas une oxygénothérapie cette disposition leur permet, vous le savez de facturer une majoration d'une valeur de 30 euros et au total jusqu'à 65 euros pour chacune des 2 premières visites par ailleurs le report de 18 mois de l'échéance de la convention médicale que vous que vous mentionnez dans votre question n'implique en aucun en aucune manière un gel de toute négociation et de tout moyen supplémentaire sur la durée du report des avancées majeures, comme par exemple l'entrée dans le droit commun de la télémédecine ou le déploiement des assistants médicaux ont ainsi été négocié depuis la signature de la dernière convention 2016 et le 8 avenants négocié à la convention de 2016 représente un investissement de 200 millions d'euros au global, enfin pour conclure, je partage et nous partageons avec vous la conviction qu'il faut continuer à améliorer l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie, de manière pérenne et non pas seulement pendant cette période de crise sanitaire, vous le savez le ministre Olivier Véran demande dans le cadre des orientations aux négociations conventionnelles pour le prochain un avenant à la convention médicale à ce qu'une attention particulière soit portée à l'accès aux soins des personnes âgées, les visites à domicile s'inscrivent bien dans cette perspective et à ce titre une majoration des visites gériatrique a été proposé par l'assurance maladie, à l'Automne 2020 représentants des médecins libéraux dans le cadre de ces négociations conventionnelles voilà monsieur le sénateur pour ces éléments de réponse. Merci monsieur le secrétaire d'État, chers collègues vous reste 30 secondes. Oui, mais merci, monsieur le ministre, si j'ai bien compris, il y a une proposition qui a été fait dans l'est, au mois de septembre dernier, mais est-ce qu'il y a une acceptation de la part du ministère ou de la sécurité sociale de revaloriser ces visites, c'était un peu la question que je posais parce que c'est une inquiétude qui est quand même forte, vu le lait, les obligations qu'ont les médecins généralistes lorsqu'ils vont à domicile, de s'équiper chaque fois avec Anne de du du matériel de protection pour justement aller voir ses malades qui sont stabilisés mais qui ne sont pas guéri du Covid, j'espère en tout cas qu'on pourra leur apporter une réponse rapidement dans le cas des discussions avec la sécurité sociale et que vous appuierez en tout cas les demandes de ses médecins généralistes qui aujourd'hui sont en grande difficulté et n'en peuvent plus, merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Laurence Garnier au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaitais attirer votre attention sur le projet de déménagement du CHU de Nantes, un projet qui est chiffré aujourd'hui a un milliard d'euros, et qui accumule les incohérences, la première d'entre elles étant la suppression annoncée de 231 l'idée est de 400 postes, vous savez comme moi que la population de Loire-Atlantique continue à augmenter et que l'enjeu du nombre de lits est tout à fait primordial la crise sanitaire, nous le montre tous les jours. Alors, vous le savez, tellement bien monsieur le ministre, que votre ministre de la Santé a annoncé au mois d'avril dernier, la révision de tous les projets de restructuration des hôpitaux, j'attends donc qu'il s'intéresse de très près au projet nantais parce qu'au-delà de ces incohérences il y a une une incohérence supplémentaires qui concerne le choix retenu pour ce déménagement, le site de l'île de Nantes, qui est un site exigu, coincé entre les 2 bras de la Loire, ce qui en fait à la fois un lieu inondable avec des surcoûts colossaux pour les travaux, un lieu très difficilement accessibles puisque, quelle que soit l'endroit d'où l'on vient, il faut franchir des ponts pour s'y rendre et puis également un lieu trop petit, puisque les surfaces réservées actuellement sont que 4 fois inférieur aux surfaces actuellement occupée par les hôpitaux nantais alors l'origine du projet c'était la volonté de regrouper les 3 sites hospitaliers nantais sur un même site, sur l'île de Nantes et on a appris la semaine dernière que compte tenu de cette exiguïté, les 3 sites existants poursuivraient leurs activités dans les années à venir. On s'apprête donc à dépenser un milliard d'euros pour avoir moins de lits, moins de postes et un financement extrêmement fragile du projet précisément conditionnée à cette suppression de lits et de comme l'a souligné récemment, la chambre régionale des comptes, monsieur le ministre, je crois que sur ce projet, nous allons tout droit au scandale sanitaire n'en soyez pas la caution, beaucoup de maires d'élus d'acteurs locaux de Loire-Atlantique sont mobilisés aujourd'hui contre ce projet, d'autres solutions existent, je compte donc sur votre bon sens pour remettre à plat ce dossier et pouvez-vous dès aujourd'hui nous confirmer que ce projet d'hôpital nantais et bien concernés par le moratoire annoncé en avril dernier par le ministère de la Santé. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci madame la la présidente, madame la sénatrice Laurence Garnier je ai développer une une vision sensiblement différente de celle que vous venez d'exposer, de partager avec nous rappeler que ce projet de de du CHU de Nantes est le fruit de 2 longues années de réflexion et de concertation ne sort pas de de terre comme ça, il a été conçu sur la base des principes d'évolutivité de modules la vérité également qui doivent lui permettent de s'adapter aux besoins et aux nouvelles pratiques et les premiers enseignements de la crise sanitaire que nous nous traversons montrent démontre que son dimensionnement spécialisé nécessaire dans un contexte de crise et pertinent, son organisation également architectural emplo apparaît également adapté à une prise en charge en contexte épidémique telle que nous le le vivons actuellement alors la crise sanitaire a démontré l'importance du maillage territorial de notre système de santé aussi, si des adaptations de cibles capacitaires devait être décliné sur le territoire de Loire-Atlantique et ce regard de l'évolution des besoins de la démographie aussi, il est essentiel qu'elles puissent avoir une traduction opérationnelle à échelle du territoire et non à l'échelle du seul projet Île de Nantes, il s'agit de pouvoir favoriser fluidifier évidemment les logiques de parcours de santé et ce, en concertation évidemment là aussi avec les élus et les professionnels de santé, alors le choix de la centralité de ce projet sur l'île de Nantes n'est pas remis en question et a au contraire été confortée lors de l'instruction du permis de construire et de l'autorisation unique environnementales qui ont été menées, le CHU de Nantes connaît une situation par ailleurs financière solide. Certifiés sans réserve et qui lui permet aujourd'hui de soutenir des investissements chambre régionale des comptes dans son rapport 2019 témoigne d'une analyse très abouti, la gestion de l'établissement et de sa dynamique de fonctionnement, elle souligne de bons résultats en état d'avancement, conforme aux attentes, ainsi que la qualité du pilotage du du projet, la situation du CHU en matière de ressources humaines et notamment d'absentéisme se situe dans la moyenne nationale, des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail sont déployés par la direction générale et l'organisation actuelle sur 2 sites de court séjour, ainsi que la vétusté, l'inadéquation des locaux sont une contrainte pour les équipes, à laquelle le projet Île de Nantes va apporter une véritable réponse et en cela, il l'emporte, nous semble-t-il, de ce que l'on en selle l'adhésion des personnels du du CHU eux-mêmes gouvernement soit convaincu, madame la sénatrice portera une attention particulière à ce que le projet puisse se mettre en oeuvre en préservant, vous avez raison, la santé financière de l'établissement et un niveau de ressources humaines qui soit adapté aux enjeux de prise en charge qui découle des nouvelles orientations telles qu'elles sont sorties du Ségur de la santé, voilà madame la sénatrice les éléments que je vous pouvez vous ce matin de la part du ministère des solidarités sont. Merci Monsieur le secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Sébastien Meurant au ministre des solidarités et de la famille. Merci madame la présidente, madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte également sur la fermeture d'un hôpital, cette fois dans le Val d'Oise, il s'agit de l'hôpital Roger Prévôt située à moi celle l'établissement 200 lit va être délocalisée, entre 2000 22 et 2024 pour être intégré au centre hospitalier de Nanterre contre la volonté des élus locaux et du personnel hospitalier des 2 structures, d'un côté, Patrick Jarry, président de l'hôpital de Nanterre et maire de la ville, juge disproportionnée cette délocalisation qui ne permettra pas, et, et, je le cite, une prise en charge digne et humaine des patients. De l'autre côté le personnel hospitalier de ce même hôpital partage ce point de vue et s'inquiète de la disparition des services dits rentables nous pneumologie réanimation chirurgie et de la culmination de structures médicales et sociales peu valorisante au sein de locaux, de plus en plus vétustes, monsieur le Ministre, comment expliquer cette logique de paupérisation de l'offre de soins à la fois dans le 95 et si j'ai un coûteux dans le 92, pourquoi ne pas faire preuve de bon sens, écoutez les élus locaux et les personnels hospitaliers qui vit ses sujets au quotidien la logique de fermer les lits d'hôpitaux et de réduire l'offre de soins pour faire des économies dans un contexte général d'augmentation et de vieillissement de la population française est tout bonnement une ineptie, le contrôleur général des lieux de privation de liberté puisqu'moi ça s'agit aussi d'un hôpital psychiatrique, mais lui met en avant, dans un rapport de visites et ont eu lieu en mai 2016 de nombreux éléments objectifs en faveur d'un maintien de cet établissement sur son territoire, Valdas Val-d'Oisien, je le cite, cadre magnifique dans un parc de 7 hectares où de nombreuses activités diversifiées permettent d'assurer la continuité des activités thérapeutiques équilibres financiers et capacité de foot d'financement dont dispose l'établissement stabilité efficacité du nombre de personnels, tous les postes sont quasiment pourvus dans des locaux adaptés aussi je vous demande si vous entendez intervenir en faveur du maintien de l'EPS Roger Prévôt ah moi celle je souhaite connaître quels moyens vous comptez dégager pour préserver les emplois des agents de l'hôpital mobilisés contre cette fermeture depuis plus de 2 ans maintenant, merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci madame la la la présidente monsieur le le sénateur Sébastien Meurant.

2020 structures ambulatoires sont déjà toutes situées dans les, dans les Hauts-de-Seine, alors, cette opération vise tout d'abord à rapprocher les lieux d'hospitalisation des lieux de vie des patients l'hôpital Roger Prévôt est en effet dédiée aux patients, aux patients du nord des Hauts-de-Seine. Il dessert pourtant une population dont il est géographiquement éloigné la recoller relocalisation pardon facilitera le maintien des Liens, des patients hospitalisés avec leurs proches et avec leur environnement, elle vise ensuite à adapter les locaux objectif du projet médical commun ce projet médical vise à favoriser les prises en charge en ambulatoire et les parcours de soins, la localisation des lits d'hospitalisation complète dans un bâtiment 9 permettra de proposer aux patients une qualité hôtelière améliorée et harmonisée cette nouvelle implantation permettra enfin le développement d'activités nouvelles, à la fois pour les jeunes adultes ou pour les personnes âgées, enfin 3ème Point. L'opération devra favoriser les Liens avec la cité, le site de moi celle a mis en place en intra-hospitalier une organisation performante et largement salué, je crois, pour proposer des activités thérapeutiques, la relocalisation au CLSH permettra de capitaliser sur cette expertise acquise pour y ajouter une dimension de lien avec l'extérieur. Ce projet consolidera les axes d'excellence du CLSH s'agisse des filières médicale, gynécologie obstétrique, ce sont des personnes âgées, l'offre destinée aux personnes en situation de précarité, il y a aussi porteur de développement de l'offre de soins en cardiologie en pneumologie en gastro-entérologie, en psychogériatrie parmi d'autres, sa mise en a fait l'objet d'une gouvernance spécifique, elle doit permettre une large concertation. Il a reçu un accueil très favorable des élus locaux des communes des Hauts-de-Seine, dont les allemand concitoyens sont actuellement, je le rappelle, hospitalisé, très loin de leur domicile lors d'un comité des élus qui a été installé le 22 janvier 2020, un accompagnement spécifique des personnels et mis en place depuis 2 ans, c'est un des volets de votre question parce qu'il y a des inquiétudes qui se sont manifestés à cet égard, des réflexions sont en cours entre les élus locaux, par ailleurs, 2 mois celle et date Hinwil pour envisager l'avenir du site lui- même, dans le respect des projets qui sont portés par chacune des communes, voilà monsieur le sénateur, les éléments, je pouvais partager avec vous ce matin. Chers collègues, il vous reste une quinzaine de secondes, si vous le souhaitez, répond. Ce secrétaire d'État, pas complètement assurée par vos propos concernant notamment le site de moi c'est ta ville où j'ai également reçu les élus locaux et je n'ai pas la même vision de Dieu que vous plus généralement dans le Val d'Oise et très rapidement, nous assistons à la fermeture d'hôpitaux

vous remercie l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Franck Montaugé au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État à la direction du centre hospitalier de Côte-d Or a soumis à la jeune se Régionale de Santé Occitanie, une demande d'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, cette demande ne s'est soldée par un avis négatif des instances décisionnaires a motivé par le choix d'installer une IRM à Auch, dans le même département, au regard des réalités de terrain cette justification ne paraît pas recevable, le centre hospitalier de et celui d'Auch ne peuvent être considérées comme concurrent ces 2 établissements contribuent conjointement à l'accès aux soins sur un territoire très affectés par la désertification médicale la raréfaction de certaines pas praticiens une population âgée et dépendante et des temps de trajets souvent longs la demande et d'équipement du centre hospitalier de Côte-d Or ne doit pas être considérée comme un luxe, elle répond à un réel besoin dans un territoire où la population vulnérable subit des inégalités très fortes en matière d'accès aux soins de santé, l'implantation d'un IRM contribuerait de plus au confortement du centre hospitalier de Cognos ainsi qu'à son dynamisme et il insufflera un nouvel élan avait le recrutement de spécialistes, il est essentiel de renforcer, de telles entités sur notre territoire national, la gestion de la pandémie de la COVID 19 a prouvé combien le maillage était des établissements mais vital dans le cas du délestage imposée par la crise sanitaire aussi je vous sollicite, monsieur le Ministre, pour que la demande du centre hospitalier de Countdown soient réexaminées dans son contexte, au regard des caractéristiques de la population qu'il sert et des difficultés d'accès aux soins de plus dans une approche d'économies de fonctionnement, relatives notamment aux transports sanitaires de cohésion et de lutte contre le renoncement aux soins cette demande d'investissement me paraît légitime et mérite d'être à nouveau étudié. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. La la présidente, monsieur le sénateur Franck Montaugé vous par votre question, la tension sur le dossier de cette demande d'implantation d'un IRM, déposée par le centre hospitalier de condom. Demande qui a été déposée durant la période de dépôt de demande d'autorisation ouverte par l'ARS Occitanie pour un scanner, un appareil d'IRM entre juin et août dernier en parallèle une autre demande d'implantation d'un IRM concernant le Centre suisse d'Ocha, avait été mise, vous l'avez évoqué dans votre question, et c'est ce dernier établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel appartient aussi le centre hospitalier de condom, qui ne dispose pas d'équipements matériels lourds en propre, rappelons que les possibilités d'autorisation en ml en Occitanie qui ont été fixées dans le schéma régional de santé pour 2018, 2022 répondre en priorité à 2 objectifs de santé pour ce volet imagerie : d'une part, prioriser les nouvelles attributions selon leur adossement à des activités fortement demandeuses d'imagerie en particulier l'activité de soins de médecine d'urgence, l'activité de neurologie et de cancérologie et d'autre part favoriser pour les nouvelles implantations la Constitution ou le renforcement de plateaux qui soit complet et diversifié, alors les possibilités d'autorisations d'implantations nouvelles d'appareils d'imagerie en Coupe n'avait pas été inscrite dans le SRS pour le Gers, elles l'ont été dans le cadre d'un besoin exceptionnel dont l'objectif était de sécuriser le fonctionnement des EMS du département suite à des difficultés majeures de gouvernance du groupement d'intérêt public en assurant la gestion jusqu'à présent, rappelons que ce GIE gère pour le compte du centre hospitalier de gauche de la clinique de Gascogne et d'un groupement de radiologues libéraux, le seul IRM qui était installés sur la ville d'Auch, dont l'activité est à plus des 2 tiers de nature privée. Il était nécessaire et urgent de sécuriser l'accès aux examens d'IRM de la population du département et l'IRM qui sera implanté dans le Gers aura vocation à desservir évidemment toute sa population et devra répondre aux besoins de maillage territorial en tenant compte des URL en en limite de ce département également. La commission spécialisée pour l'organisation des soins de la région Occitanie a donné un avis fortement favorable à l'installation de l'IRM au centre hospitalier de gauche comparativement à celui donné pour le le centre hospitalier de de condom, le DG, directeur général, pardon, de l'Agence Régionale de Santé à noter l'activité importante et pertinente du scanners installés au CH de condom, dont la place et le rôle sur son territoire, sont bien connues et rendra sa décision au plus tard le 22 mai par ailleurs conformément à ses engagements auprès des fédérations et suite à l'initiative de la conférence régionale de la santé de l'autonomie, les travaux de révision du volet imagerie du SRS ont débuté en juillet 2020, associant notamment radiologues et cliniciens ces travaux doivent aboutir à la formulation de nouveaux besoins Duhamel pour la région Occitanie courant 2021 et à la définition de nouveaux objectifs d'implantation de par département, je conclus vraiment, excusez-moi, madame la présidente, pour vous dire, Monsieur le Sénateur, que la réforme des autorisations d'activités de soins en cours dans le cas de ma santé 2022 s'attache également concernant l'imagerie à simplifier l'ajustement de la réponse aux besoins via une réflexion sur un assouplissement du régime actuel, voilà monsieur. Merci monsieur le secrétaire d'État, vous savez, chers collègues, 45 secondes. Et merci monsieur, monsieur

à condom fragilise le le territoire de santé, donc effectivement le centre hospitalier d'Auch et le l'établissement support on habitue les gens aller à Agen et caetera et et je pense que dans une optique de réponse

ça a été le cas aussi de la direction de l'hôpital de de de Caunes et aujourd'hui voilà, ils sont, ils sont très déçus, je termine sur un point qui est relatif à la démographie médicale, la démographie, les midi peu elle dépend aussi de la qualité des équipements et des actes que l'on peut réaliser au au sein des centres hospitaliers et c'est typiquement le cas pour la problématique du du du de monde. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Patrice Joly au ministre des solidarités et de la santé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite vous relayer les inquiétudes Monsieur le Ministre, des représentants des grandes organisations et fédérations de l'aide à domicile, concernant le calendrier incertain du projet de loi relatif au grand âge et à l'autonomie, comment, pour commencer, ne pas rappeler la forte mobilisation des acteurs accompagnant les personnes âgées, le 30 janvier 2018 pour exprimer leur malaise, ce fut leur manière de dénoncer les moyens humains et financiers, manquant ainsi que les effets délétères de la réforme de la tarification de 2015 depuis un rapport portant plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge, avec plus de 175 propositions pour refonder la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie a été remis en mars 2019 la mission sur l'attractivité des métiers du grand âge et de l'autonomie, quant à elle, a rendu ses conclusions en octobre 2019 ces 2 rapports ont été ont ont mis en exergue la nécessité d'avoir une réflexion la réelle relatives aux métiers du comptage leur qualification diplôme stature rémunération ainsi que conformation préparant à ces métiers, vous le savez, Monsieur le Ministre, les directeurs d'Epad ont des difficultés à recruter des personnels qualifiés et se retrouve à embaucher des encadrants non diplômés mais qui apprennent un métier sur le terrain, donc sans formation théorique, et sans obtenir la qualification professionnelle reconnu ces employées, majoritairement des femmes se retrouve cantonné sur des postes à faible rémunération sans Policy pas sans possibilité d'évolution rendant peu attractifs ces emplois, monsieur le Ministre, les enjeux sont cruciaux et connue de tous. La problématique de la population vieillissante devient plus aiguë en raison de l'entrée des baby-boomer, dans les âges avancés, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées se pose avec une plus grande acuité, 3 ans après le mouvement social d'ampleur dans les établissements et les services d'aide à domicile pour personnes âgées, les professionnels restent très inquiets et sont à l'attente de la mise en oeuvre de mesures concrètes d'un calendrier stable et d'une réforme lisible, coordonner et financer une loi a été annoncée à l'Automne 2000 19 et désormais repoussé éventuellement à l'été 2021, selon la ministre madame bourguignon le président Emmanuel Macron ne l'a d'ailleurs pas mentionné parmi ses priorités lors de ses voeux du 31 décembre dernier ce qui est surprenant, aussi je souhaite connaître les intentions du gouvernement en la matière, je vous remercie. Si Madame la la présidente monsieur le monsieur le sénateur Patrice Joly, vous m'interrogez sur le calendrier gouvernemental en matière de prévention et de soutien à l'autonomie au grand âge, calendrier, vous le connaissez, il a déjà débuté, il est bien entamée, de nombreuses concertations sont déjà tenus sur des questions organisationnelles avec le rapport sur sur le renforcement de l'attractivité des métiers du grand âge avec le rapport de de Myriam El Khomri et de nombreuses autres ces rapports, ils ont eu 2 premières traductions en attendant la réforme globale sur laquelle nous travaillons dont le projet de loi grand âge et autonomie, qui sera examiné dès que nous aurons surmonté la crise sanitaire que nous traversons, c'est dans cet esprit qu'ont été adoptés, d'une part, la loi relative à la dette sociale à l'autonomie, ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 qui contenait un certain nombre de de dispositions, il y a déjà eu des avancées majeures, premières d'entre elles étant la création de cette 5ème, branche de la Sécurité sociale avec la protection du risque de perte d'autonomie, c'est une première étape essentielle pour la concrétisation de notre ambition à la matière évidemment ne s'arrête pas là le défi démographique Basson bat son plein et nous avons à coeur de faire vivre de nouvelles solidarités pour leur donner corps, il nous faut repenser l'accueil de nos concitoyens, en perte d'autonomie, il le demande un répondre à leur attente de mieux vivre chez eux ou dans un établissement qui sont en phase avec leurs aspirations pour cela, il faut à la fois des lieux adaptés et des personnes pour y travailler, nous avons oeuvré sur ces 2 sujets, le plan de relance d'une part, vient financer la rénovation de près de 30000 places en établissements de Ségur de la Santé vient quant à lui, rehaussé le salaire des professionnels en pas, d'un montant minimum de 160 à 181 5 euros Net par mois, les professionnels du domicile ne sont pas en reste le point d'indice a enfin été dégelés, le gouvernement a décidé d'accompagner le financement de la revalorisation des salaires, des aides à domicile qui dépendent normalement des seuls départements, vous le savez, 200 millions d'euros sont ainsi mobilisés chaque année par l'État, en plus de ce que les conseils départementaux mobiliseront eux- mêmes et Besançon évidemment majeur la crise les a mis en relief un peu plus encore, elle mobilise, vous vous en doutez bien pleinement Olivier Véran et et Brigitte bourguignon, qui travaille à la fois activement sur la protection de nos aînés, face à la crise sanitaire et sur le projet de soutien à l'autonomie que nous développons et notre priorité est de faire face à la crise, mais nous continuerons et nous continuons de porter notre ambition par tous les moyens, tant que celle-ci ne sera pas pleinement juguler voilà monsieur le sénateur pour ces éléments de réponse. Merci monsieur le secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Christine Herzog transmises au ministre des solidarités et de la santé. Ma question s'adresse à Madame la ministre des collectivités territoriales, sur le rôle et les responsabilités des maires de la gestion actuelle de la pandémie de Covid 19 et de la vaccination. Monsieur le ministre, la Moselle a été durement touché par la crise sanitaire du COVID 19 avec 1490 décès depuis mars, soit 22 % du Grand-Est et les élus ont dû faire face malgré leur manque de moyens à des situations difficiles. Les premiers ministres qui se sont succédés depuis mars 2020 assurer au Sénat il y a la ville de Metz, que l'État, mené des actions ciblées de prévention de l'épidémie d'assistance et de gestion de la vaccination et qu'ils avaient désormais les moyens de contenir la contamination lorsque les clusters sont identifiés, notamment pour la dernière souche appelée variant les chiffres cependant ne baissent pas au contraire au 17 janvier nous avons 204 nouveaux cas pour 100000 habitants en Moselle, alors que la moyenne nationale est de 188. Le maire en tant qu'élu et 1er magistrat de sa commune et la personne de confiance vers qui nous les concitoyens se tourne en cas de difficulté car le maire est le mieux placé pour la vaccination, il n'y a pas, il n'a pas été sollicité, sauf pour les grandes métropoles c'est étonnant d'ailleurs, car le maire peut influer grandement sur la décision de ça de la de de faire vacciner. Plus d'un 1000000 d'Allemands ont été vaccinés contre 422000 Français et plus de 100000 dans les régions, frontalier de la Moselle, contre 39000 pour le grand test, nous sommes très très en retard, vacciner les personnes âgées, est une bonne chose, les vacciner ceux et celles qui sont associés à ces personnes est indispensable pour éviter la contamination, afin de ne pas aggraver la crise économique, il faut aller plus vite et vacciner davantage actif. Je souhaite donc savoir quels sont les moyens mis à disposition des élus locaux et quels seront leurs rôles et responsabilités dans les actions des prochaines vaccinations et du passeport vaccinal, par ailleurs, dans l'éventualité où l'école serait touchée par un nouveau confinement, je vous demande de préciser quand et comment le gouvernement envisage d'associer les maires au protocole sanitaire à mettre en place pour les enfants. Je vous remercie, Peut être plus clair, c'est la conviction qui est la nôtre, la concertation et quotidienne au niveau local avec les préfets avec les agences régionales de santé dans le département de la Moselle, 2 instances de concertation, vous le savez, se réunissent à une fréquence hebdomadaire au niveau stratégique, il s'agit du collègue sous le pilotage du préfet qui réunit tous les parlementaires du département compris vous je je pense le président de la région Grand-Est, les élus des grandes villes mais aussi 3 représentants des maires ruraux au niveau opérationnel, nous avons instituée par instruction ministérielle datée du 15 décembre dernier une cellule départementale de vaccination sous la coprésidence du préfet du département et de la directrice générale de l'ARS et qui réunit l'ensemble des parties prenantes des mères en font partie, depuis la fin décembre, par l'intermédiaire des cellules départementales de vaccination, nous avons demandé au maire de proposer des lieux adaptés à l'ouverture de sondes vaccinaux et de prendre attache auprès des personnes vulnérables, concernés par cette nouvelle étape de vaccination qui s'est ouverte lundi dernier, je tiens à les remercier, à l'occasion de votre question, d'avoir contribué par leur expertise au plus près du terrain, la création, à l'ouverture de plus de 800 Centre à ce jour, nous savons pouvoir leur faire confiance dans la mobilisation des acteurs des territoires pour l'organisation de la vaccination malgré des contraintes logistiques forte qui s'impose à nous tous, et nous continuons dans ce sens en les associant avec le ministère de l'Éducation nationale au protocole sanitaire mises en Oeuvres dans les établissements scolaires pour garantir leur ouverture depuis la rentrée, ce protocole sanitaire et renforcé, vous l'avez évoqué pour éviter le brassage entre les classes, les activités physiques et sportives scolaires en intérieur sont suspendus et nous décuplant notre capacité de dépistage dans les écoles avec un objectif de 300000 tests par semaine, le rôle des maires sera aussi 1er dans le transport des personnes vers les cendres de vaccination, ministre des solidarités, de la santé, a eu l'occasion d'échanger à ce propos avec le président de l'AMF pour réaffirmer le le principe la stratégie vaccinale française repose sur les connaissances scientifiques dont nous disposons et sur les recommandations de la Haute autorité de santé, vous le savez depuis le démarrage de la campagne vaccinale, nous avons été transparents sur les approvisionnements, nous avons transmis aux élus locaux, via les associations d'élus, les préfets, les directeurs généraux d'ARS, les nombres de vaccins, les lieux et les dates de livraison dans les établissements pivot. 17 janvier, plus de 422000 personnes avaient pu recevoir une première injection du vaccin dans notre pays environ 1,6 millions de doses ont été livrées, auxquels s'ajouteront 315000 doses Pfizer supplémentaires d'ici le 20 janvier nous avons demandé aux préfets, aux ARS d'adapter l'ouverture des Centres de vaccination caractère progressif du calendrier d'approvisionnement, il est important que le dialogue puisse se tenir localement pour optimiser la vaccination en fonction des doses disponibles en organisant au mieux la coordination des horaires d'ouverture des différents centres et éviter l'éparpillement des ressources médicales et paramédicales de la question des doses dans les établissements ont été faites pour coller à la réalité des territoires aux besoins de leur population, en utilisant toutes nos ressources en vaccins, tout est fait pour éviter les stocks dormants, m'y autorisez c'est un sujet important, merci beaucoup madame la la présidente, la campagne de vaccination durera jusqu'à l'été, à mesure que les vaccins seront autorisés, livré à l'Union européenne, les volumes globaux dont nous disposons, négocier au niveau européen, vous le savez sont limitées durant ces premières semaines il faudra quelques semaines pour que l'ensemble des personnes de plus de 75 ans ou atteints de pathologies graves puissent être vaccinés, il s'agit d'une course de fond, dans laquelle l'engagement de chacun doit primer et, s'agissant enfin du guide relatif à l'organisation de la vaccination dans les Ehpad et les USL, celui-ci était à destination des directeurs d'établissements, il est le produit des interrogations légitimes de ces derniers au regard de la fragilité des publics concernés en aucun cas un frein à la vaccination, le recueil du consentement s'dans le cadre du droit et des règles en vigueur connue et pratiquée par les médecins, en vertu du Code de la santé publique et du code de déontologie, voilà madame la scène. Merci monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il vous reste en seconde, si vous souhaitez répondre. Merci beaucoup pour cette précision Monsieur le secrétaire d'État, malheureusement, c'est que des effets d'annonce, ce n'est pas une réalité du terrain, ce qu'on vous demande, soyez beaucoup plus clairs dans leur communication, vous et votre collègue va le gouvernement rassurer les gens et faites confiance aux élus, je vous remercie. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Gilbert Roger, au ministre de l'Économie, des finances et de la relance. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, j'ai attiré l'attention du ministre de l'Économie et des Finances sur la surprime appliquée par les loueurs de voitures aux jeunes conducteurs, c'est-à-dire âgés de moins de 26 ans, du fait du risque d'accident plus élevé pour cette catégorie de conducteurs, les prix varient selon les sociétés de location, mais certains loueurs pratiquent des surprimes très importantes jusqu'à 2 fois le tarif normal, par ailleurs, les sociétés de location pratique la surprime des jeunes conducteurs ne communiquent pas toujours les montants de leurs tarifs, je souhaiterais savoir si le gouvernement serait prêt à réglementer cette surprime jeune conducteur pratiqués par les sociétés de location de véhicules pour en limiter l'application aux conducteurs ayant eu au moins 2 ans de permis afin d'éviter l'application de ses tarifs prohibitifs merci. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Oui, bonjour, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gilbert Roger vous attirer l'attention du gouvernement sur les suppléments que les loueurs de voitures applique consommateurs âgés de moins de 26 ans, je rappelle que s'il est interdit de refuser ou de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition, fondée sur l'âge, rien n'interdit aux loueurs d'appliquer des suppléments ainsi le défenseur des droits, a souligné dans une décision du 16 décembre 2014 que la fourniture d'une prestation de location de voitures à des conditions tarifaires distinctes ne caractérise pas une différence de traitement prohibé, sauf si cela manifeste une volonté d'exclure les personnes concernées s'apparente alors à un refus implicite, toutefois, il est indispensable que le consommateur en soient parfaitement informés avant la conclusion du contrat des dispositions réglementaires vice dans ce cadre à protéger le consommateur en lui permettant d'avoir une connaissance précise des montants de ces suppléments avant de s'engager contractuellement ce cadre réglementaire vise à favoriser la transparence des prix au bénéfice d'une concurrence accrue et d'une modération tarifaire, les services de la DGCCRF effectue régulièrement des contrôles dans ce secteur, les agents portent une vigilance particulière à l'absence de refus de vente, il y a l'âge du consommateur et à la bonne communication des tarifs, les consommateurs peuvent, si cela est nécessaire, adresser des réclamations sur le site mis en place par le gouvernement, signal Point conso pour finir, en application de l'article L 410 2 du Code du commerce Le gouvernement peut réglementer les prix dans les secteurs où les zones où la concurrence par les prix et limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement telle n'est pas le cas pour le secteur de la location de véhicules qui se caractérise par une forte concurrence entre plusieurs sociétés dont les agences sont le plus souvent implantés dans les mêmes zones de commercialisation comme les aéroports, gares au centre-ville, ce qui permet aux consommateurs d'accéder à différentes offrent secteur se caractérise de plus par l'émergence de nouveaux canaux réservations notamment en ligne, rendant les comparaisons tarifaires plus aisée et favorisant de facto à la concurrence. Merci, chers collègues, il vous reste une minute 27 si vous souhaitez réplique. Je vais pas tenir une minute 27 mai quand même dire qu'effectivement, si on prend l'exemple des aéroports ou des gares, vous vous apercevrez mais peut-être que ni moi, ni vous ni moi n'avons maintenant cet âge de moins de 26 ans que sur ce qui concerne les surprimes elles sont équivalentes et très élevés, notamment pour les jeunes conducteurs, monsieur le ministre, ce que j'aimerais, c'est que l'on regarde très sérieusement, pas uniquement les statistiques de votre service, c'est qu'un jeune qui passe le permis aujourd'hui qui peut commencer à apprendre à conduire avant l'âge de 18 ans, à partir du 15ème 16ème année, il commence à apprendre à conduire, à 18 ans, il a permis à 20 ans il a ces fameux 2 ans permis qui font que des autorisations supplémentaires lui sont donnés et les compagnies d'assurance traditionnelle pour les voitures personnelles sont moindres et on lui laisse une surtaxation jusqu'AFSA 26ème année franchement essayer de retourner dans votre bureau tout à l'heure et de dire il y a un truc qui va pas, essayons quand même de regarder ça pour la jeunesse, durement touchée, merci. Merci, cher collègue, vous avez tenu vaut 1 minutes 27 l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Cathy à pour Sopot liée au Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des finances et de la Relance chargée des comptes publics. Merci madame la présidente, à l'heure, ma question s'adresse au ministre de l'action et des Comptes publics, monsieur le ministre, votre prédécesseur a lancé une réforme qui passe par la fin des transactions en numéraire dans les trésoreries, mais également par un bouleversement total de la présence des finances publiques dans les territoires avec la fermeture de trésorerie, or, que ce soit auprès de votre prédécesseur de vous-même, monsieur le ministre, ou de vos services, nombre de maires et d'élus de mon département, le Pas-de-Calais, ont fait part de leurs craintes mais aussi de leur colère en effet avec celte mal nommé réforme du nouveau réseau de proximité vous prétendez, améliorer la présence des services publics dans les territoires, en effet, les maires et élus voient cette réforme comme un nouveau transfert de compétences envers les collectivités territoriales, sans compensation de l'État, les accueils de proximité, les France services sont bien souvent à la charge des collectivités qui doivent assumer seul des compétences autrefois prises en charge par l'État et sans compensation monsieur le Ministre, les services publics de proximité sont essentiels, ils ont montré toute leur efficacité en cette période de crise sanitaire leur connaissance du terrain et leur implantation en proximité, en font des maillots indéniable pour la sauvegarde de nos territoires, dernièrement, le directeur du Pas-de-Calais a annoncé dans la presse que les particuliers pourraient à nouveau payer leurs amendes et factures de divers services dans les permanences municipales ou les points d'accueil de proximité alors que les paiements chez les buralistes engendre un surcoût pour l'État, pourquoi avoir mis en place cette réforme pour finalement revenir à un paiement possible auprès des agents des finances publiques, une réforme des moyens à moyens décroissants n'est pas compatible avec la réaffirmation de la République dans tous les territoires, les circonstances sanitaires ne permettent pas de tenir des réunions de travail et de concertation entre les services entre les élus et l'État et services des directions départementales et générale des finances publiques, je vous demande de bien vouloir suspendre la mise en application du nouveau réseau de proximité afin que le dialogue puisse s'engager sereinement face aux alertes des élus, des usagers et des agents qui vous envisagez ou vous envisagez la des milliers de suppressions d'emplois, je vous remercie.

je souhaite tout d'abord vous rappeler au nom d'Olivier Dussopt notamment les objectifs du nouveau réseau de proximité, proximité de la DGFIP et les caractéristiques de la mise en 9 pour le définir maillage de la DGFIP, l'un des plus denses de l'État reflète la diversité de ces missions, mais également une organisation qui ne correspond plus aux besoins actuels, le nouveau réseau de proximité vise précisément à rapprocher ça reste public de nos concitoyens et de tenir compte des besoins spécifiques de nos publics en offrant aux élus et à nos concitoyens un service modernisé, plus proche et répondant à leur demande, concrètement, il consiste à augmenter le nombre d'accueil de proximité de plus 40 % et de développer le conseil aux élus locaux, près de 1304 seront dédiés à terme à cette mission de conseil financier, fiscal, budgétaire et comptable en parallèle les activités de gestion seront mutualisés au ça au sein des services de gestion comptable, pour gagner en efficacité et en rapidité la DGFIP s'attache à mettre en place un accueil de proximité, aussi bien en France, service Cormery, notamment dans les communes les plus reculées et éloignées des centres urbains, les usagers bénéficient d'un accueil dédiés par des enjeux agents aux compétences élargies qui prendra en charge toute demande en complément, la possibilité de payer chez les buralistes agréés implanté dans les villages se déploie progressivement et offre aux usagers une facilité horaires plus larges que celles des services de la DGFIP pour définir l'organisation de ses services, la DGFIP a engagé il y a un peu plus d'un an, une démarche inédite concertée partenarial auprès des élus et de ses agents, à ce jour, au plan national des conventions départementales ont été signés dans 37 départements, avec les présidents de conseils départementaux, tout est assez souvent, ceux de l'association départementale des maires et le préfet parallèlement, plus de 400 conventions ont pu être signé avec les présidents d'EPCI au total 78 départements ont signé une charte soit départemental soit avec un EPCI le projet du nouveau réseau de proximité se construit dans le dialogue et au bénéfice des territoires ruraux qui ont tout à gagner à la nouvelle organisation de la DGFIP, qui s'adapte aux besoins de ces usagers et de ses partenaires dans le cas particulier du Pas-de-Calais, la DGFIP des 62 et présente aujourd'hui dans 42 communes à l'issue de cette réforme, elle sera implantée dans 52 communes soit une présence renforcée dans 10 communes supplémentaires, je prends merci. Merci monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il vous reste une dizaine de secondes pour jouer juste 2. De 11 secondes monsieur le ministre, vous m'excusez, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes moderne que vous êtes proche, vous êtes dans la proximité et vous supprimez alors moi il faut m'expliquer comment avec de telles suppressions, vous allez pouvoir être encore dans la proximité, je vous remercie. Merci, chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Olivier Rickman au ministre de l'Économie, des finances et de la relance. relance. La présidente, monsieur le ministre, ma question se rapproche étroitement de la question de ma collègue a pour ce Poli mais comme disait le philosophe, répété, répété, il en restera toujours quelque chose depuis 2019 les finances publiques ont engagé au niveau national, une vaste opération de réorganisation appelé INRP nouveaux réseaux de proximité, je connais partage en partie vos objectifs, aucune administration ne peut rester figés et nous devons exploiter les potentiels offerts par les nouvelles technologies. Pour autant, je souhaite également partager avec vous, le constat des maires et des conseillers départementaux de la Haute-Saône relayer leurs questions, le constat est d'ordre sociétal pour des millions de Français déjà confronté à la fracture numérique et dont les capacités sont inexistantes ou limitées en informatique cette dématérialisation à marche forcée est un accélérateur du délitement des relations humaines, leurs questions et d'ordre très pratique, elle porte sur la qualité du service rendu, par notre administration ce nouveau réseau, fait la part belle aux maisons des services au public, M. SAP et aux établissements France service or nul ne peut affirmer qu'un accueil par les employées de ces structures sera à la hauteur du service rendu par un agent de la DDE, Philippe, à titre d'exemple auprès de quelle instance de proximité, un contribuable souvent modestes pour, a-t-il argumenté afin de bénéficier d'un plan d'étalement d'une dette. Sur un autre plan qui intéresse tout particulièrement les collectivités locales, la fermeture de trésoreries de proximité fragilisera les régies municipales dès lors que tous les paiements perçus ne peuvent être matérialisée, je pense aux forains sur les marchés et au nombre insuffisant de bureaux de poste pouvant recevoir des versements. Monsieur le ministre comment entendez-vous assurer la qualité du service rendu aux administrés et quelle bornes mettrez-vous à la démarche de dématérialisation continue qui nous entraîne progressivement vers une déshumanisation et qui, de mon point de vue est insupportable. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et Madame la la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Olivier Rickman. Le maillage de la DGFIP, je le disais, l'un des plus denses de l'État reflète la diversité des missions, mais également une organisation qui ne correspond plus aux besoins actuels, vous l'avez d'ailleurs dit dans votre propos, le nouveau de réseaux de proximité vise précisément à rapprocher les services publics de nos concitoyens en ligne et hors ligne et à tenir compte des besoins spécifiques de nos différents publics en offrant à aux élus et à nos concitoyens un service modernisé, plus proche et répondant mieux à leur demande, le MRP se traduira ainsi par une augmentation du nombre d'accueil de proximité de plus de 40 % je l'ai dit en France, service en mairie, notamment dans les communes les plus reculées et éloignées des centres urbains, il s'agit donc tout particulièrement de se rapprocher des usagers les moins mobiles et les moins à l'aise avec le numérique, afin de veiller à garantir l'accès de tous à nos services, notamment dans les communes les plus éloignées des centres urbains, s'agissant de la dématérialisation la DGFIP veillent à ne pas l'imposer à ses usagers à cet égard la déclaration en ligne n'est d'ailleurs, je le rappelle obligatoire que pour ceux qui ont sont en capacité de la réaliser et services en ligne et les services téléphoniques, tout comme les échanges en visioconférence qui commencent à être proposés proposés donc en complément et non au remplacement des accueils physiques, ils répondent à une attente très forte d'ailleurs d'une grande partie de du droit, en majorité des usagers qu'il faut également prendre en compte et qui souhaitent lorsque c'est possible, réaliser leur démarche en toute autonomie ou être assisté à distance afin d'éviter de se déplacer, par ailleurs, afin d'un compagnon, les usagers qui le désirent dans leurs premières démarches en ligne la DGFIP met à leur disposition dans le Hall de ses cendres des finances publiques, mais aussi dans les relais externes, notamment les structures France, service des ordinateurs et une offre d'accompagnement pédagogique, l'enjeu est donc de permettre à chacun d'utiliser les différents canaux de contact proposé en favorisant l'autonomie mais en accompagnant et en renforçant en parallèle la présence de proximité s'agissant de la qualité du service offert dans les accueils de proximité, la DGFIP, il porte une grande attention aussi bien dans les francs service que pour ses permanences en mairie, il convient de rappeler que les structures France services doivent répondre à des critères exigeants pour obtenir ce Label et que tous leurs animateurs suivent un cycle de formation très complet, les usagers bénéficient ainsi d'un accueil dédiés par des agents aux compétences élargies qui prennent en charge toute demande de 1er niveau et tous souhaitent d'accompagnement dans la réalisation d'une démarche qu'elle soit réalisé sur papier ou en ligne, par ailleurs, pour les questions plus complexes, les agents des finances publiques seront disponibles pour y répondre, soit à distance soit lors des permanences organisées notamment, mais enfin la DGFIP s'était engagé à assurer conjointement avec les élus, un suivi de cette nouvelle organisation pour s'assurer que celle-ci répond bien aux usagers et aux attentes des élus en complément, je le rappelle, la possibilité de payer chez les buralistes agréés implanté dans les villages se déploie progressivement et offre aux usagers une amplitude horaire plus large que celle des services de la DGFIP, je vous remercie. Merci monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, vous avez 27 secondes pour répondre et si vous le souhaitez. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Ne vous faites pas d'illusions, ces restructurations et fermetures de services éloigne toujours plus les usagers des services de la DGFIP. Ne niait pas l'évidence : il faut que le gouvernement rompe avec l'hypocrisie et assume le fait que la fermeture des trésoreries provoquera un affaiblissement de la qualité de l'accueil et du conseil fiscal il accentuera inexorablement le sentiment d'abandon bien légitime par l'état de nos territoires ruraux, la France n'est pas uniforme, Monsieur le Ministre, vous semblez l'oublier. Merci, merci, chers collègue lors du jour appelle la question orale de monsieur Jean-Yves Roux à la Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des finances et de la Relance chargée de l'industrie. Merci madame la présidente, je dois vous dire en préambule, combien je regrette que ministre s'occupe indirectement de ce dossier majeur ne soient pas présents aujourd'hui pour répondre à ma question, monsieur le ministre, avec 30 centrales hydroélectriques et 17 barrages répartis dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, notre région contribue à la bonne santé de l'hydroélectricité en France seconde source d'énergie renouvelable en France, or depuis 2020, l'entreprise EDF Hydro-Méditerranée qui assure l'exploitation des principaux aménagements hydroélectriques est en cours de réorganisation, il est tout d'abord prévu de rattacher 85 agents installé dans l'arrière-pays niçois et sur les aménagements de l'Argentière dans Hautes-Alpes à une unité nationale hydraulique, basé à Lyon, par ailleurs, EDF Hydro-Méditerranée prévoit dès l'été 2021, une restructuration de son siège marseillais, ainsi que des entités d'Aix-Marseille de Sainte-Tulle près de la gare d'Aix-en-Provence TGV, ce projet de restructuration, il faut le souligner, entraînera une perte d'emploi sur Marseille, mais aussi sur le site florissante de Sainte-Tulle dans les Alpes-de-Haute-Provence, de plus, le Centre conduite hydroélectrique de l'aménagement Durance Verdon sera lui aussi transféré à Lyon et, ce qui contribuera encore à détruire 12 emplois Directs sur le site de Sainte-Tulle, monsieur le ministre, le Centre conduite hydroélectrique, assure un rôle majeur dans la synchronisation des 18 centrales hydroélectriques permettant un transfert d'eau instantané de ces repensant vers l'étang de Berre cet aménagement et, de fait, indispensable, la sécurisation du système électrique région sud de même lors du passage de crue, le site permet de garantir la sécurité des personnes et des biens, depuis sa création en 1981 le Centre conduite hydroélectrique de Sainte-Tulle engendrer des aménagements multi- usages très divers, depuis l'hydroélectricité, la fourniture d'eau potable, l'irrigation et bien sûr les activités de tourisme indispensables à l'écosystème de notre département, monsieur le Ministre, pour nous, la gestion optimale des centrales hydroélectriques ne passe pas par les activités à la coupe aussi, pouvez-vous nous donner des garanties sur l'avenir du site hydroélectrique des Alpes-de-Haute-Provence, quelle position défend l'État et le gouvernement pour préserver ces aménagements et éviter tout démantèlement délocalisation il y à terme une privatisation de la gestion partagée de nos barrages et de la ressource en eau, car nous nous en voulons pas, je vous remercie. mesdames et messieurs les sénateurs, pardon monsieur le sénateur Jean-Yves Roux je vais d'abord excuser l'absence de mes collègues, Barbara Pompili et Agnès Pannier Runacher pour répondre à ces votre question sur les projets de restructuration d'EDF Hydro-Méditerranée qui concerne particulièrement le site de Sainte-Tulle l'aménagement de la Durance et du Verdon est unique en France, représentant une puissance de 2000 mégawatts la production hydroélectriques jouent un rôle essentiel pour le système électrique régional en représentant 50 % de la production régionale mais aussi pour les usages multiples de l'eau comme le irrigation l'eau potable, l'eau industrielle ou encore le tourisme elle engendre ainsi des retombées économiques importantes sur votre département, je sais qui me tiennent à coeur, avec 3,6 millions d'euros d'achat locaux en 2000 19 et 26 millions euros d'euros d'impôts locaux et de taxes en 2018, un projet de réorganisation visant à moderniser les outils de pilotage des centrales hydrauliques d'EDF est en effet envisagé, vous l'avez évoqué celui-ci aurait un impact très limité sur la présence des salariés d'EDF sur le territoire, salariés qui se comptent par centaines pour la totalité de l'aménagement Durance Verdon ne concernant pas les ouvrages d'EDF à proprement parler, les barrages, les usines et les ateliers, le projet n'droit d'ailleurs, au demeurant pas d'impact sur les achats locaux ni sur les retombées fiscales en lien avec l'activité industrielle d'EDF, toutefois, le projet de réorganisation concerne bien 25 salariés actuels du site de Sainte-Tulle qui seront désormais rattachés à l'État-Major de l'unité actuellement répartis sur 3 sites : Marseille, Aix-en-Provence et Sainte-Tulle mais qui sera regroupée courant 2021, à Aix-en-Provence, c'est 25 25 salariés pourront travailler à distance plusieurs jours par semaine, soit depuis lors de l'de l'ordre à leur domicile, pardon en télétravail soit depuis le site de Sainte-Tulle ces salariés et leurs familles, attaché aux territoires et à son cadre de vie pour donc demeurer enfin à l'horizon 2022 2025 10 salariés en charge de la télé, conduite des aménagements sont concernés par la Constitution à Lyon d'un pôle national dans le cas du projet de modernisation, tu peux l'otage des centrales hydrauliques pour répondre aux évolutions du marché ou au nouveau code de réseaux européens, il leur sera proposé soit de rejoindre à Lyon de leur activité actuelle soit de poursuivent leur parcours professionnel, sur d'autres activités sur la Durance voir dans d'autres entités du groupe EDF, pour ceux qui le souhaiteraient, soit ils assuré, Monsieur le Sénateur, que nous suivons avec la plus grande attention ce projet de restructuration et que nous sommes vigilants, vigilant, pardon à ceux que l'activité hydroélectrique demeurent sur votre territoire, je vous remercie. Merci monsieur le secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Michel Canevet au ministre de l'Économie et des finances et de la relance. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, monsieur le ministre, vous étiez dans le centre Finistère, voilà une dizaine de jours, vous étiez à Varennes sur Allier ce week-end, vous avez pu vous rendre compte de l'importance de l'agriculture dans les zones rurales, agriculture, vous avez pu vous en rendre compte, aussi, qui souffre terriblement, pour un certain nombre de productions, je pense en particulier aux productions bovines et aux productions des tiers puisque les producteurs ont du mal à gagner leur vie, de par la vente de leurs produits, on espère bien sûr une évolution technologique, notamment le recours aux outils connectés, bien entendu, pour améliorer la productivité, mais cela ne suffira pas vous vous rendez compte par ailleurs que dans notre pays, hé bien, la grande distribution est concentré entre quelques mains et concentre l'essentiel des ventes des produits, le gouvernement a présenté au Parlement, la proposition de loi qui fut votée en en 2018, mais qui n'a pas apporté des réponses à l'ensemble des problématiques auxquelles les producteurs se sont affrontés, et notamment à la possibilité de pouvoir gagner leur vie, de par le fruit de leur travail il faut s'atteler à d'autres axes de travail maintenant pour pouvoir dégager des solutions aux États-Unis en 1000 depuis 1936 il y a le Robinson, pas de Man Act, est un dispositif qui oblige les PME à vendre au même prix à l'ensemble des distributeurs, la production de façon à éviter la pression par les volumes, pouvez-vous m'indiquer monsieur le ministre, si le gouvernement peut envisager des solutions permettant enfin à l'ensemble des producteurs de gagner leur vie par le le la vente de leurs produits. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Michel Canevet, le gouvernement est pleinement engagé dans la lutte conte les pratiques commerciales déloyales, vous l'avez rappelé en 2018, le président de la République a lancé les états généraux de l'alimentation, processus de concertation réunissant l'ensemble des acteurs de la filière qui a abouti au vote de la loi dite également, il faut souligner opaque, auparavant, le législateur a multiplié ses interventions dans le domaine des relations commerciales loi Galland 1995 loi sur les nouvelles régulations économiques en 2001 loi en faveur des petites et moyennes entreprises loi Dutreil en 2005, loi de modernisation de l'économie en 2008 loi Hamon en 2014 loi Sapin II en 2016 aujourd'hui, il importe de laisser les mesures Egalim produire leurs effets, d'autant qu'il est encore trop tôt pour mesurer leur impact notamment sur le revenu des agriculteurs, c'est pour cette raison que le Parlement, par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique adopté en octobre dernier a prolongé jusqu'en 2023 l'expérimentation des mesures d'encadrement des promotions et de relèvement du seuil de revente à perte par ailleurs les interprofessions commencent à élaborer leurs indicateurs de coûts de production, comme le prévoit la loi, notamment dans la filière laitière que vous citiez, il est nécessaire de laisser le temps aux opérateurs de s'emparer du texte et de les inciter à la contractualisation à l'amont dans les filières et la DGCCRF par son programme de contrôle les pousse en ce sens il n'apparaît donc pas opportun au gouvernement de légiférer à nouveau à court terme, notamment pour instituer une mesure rétablir l'interdiction de discrimination abusive, qui a été supprimée par le législateur en 2008, je vous le rappelle, vous évoquiez également la possibilité de poursuivre les distributeurs sur le fondement du déséquilibre significatif, je vous informe que le ministre chargé de l'économie assigne régulièrement le distributeur devant les tribunaux de commerce pour des pratiques abusives envers leurs fournisseurs depuis 2008 de nombreuses décisions de justice ont été rendues dans des affaires initiées par le ministre ainsi 16 millions d'euros d'amende civiles ont été prononcées contre les auteurs de telles pratiques parfois également condamné à restituer aux fournisseurs lésés, plus de 180 millions d'euros indûment perçus très récemment, Bruno Le Maire a engagé 2 actions judiciaires dans lequel il demande au juge la condamnation à près de 220 millions d'euros d'amende civile en 2020, il a développé le recours aux sanctions administratives dans le domaine de pratiques restrictives de concurrence en sanctionnant 4 grands opérateurs de la distribution alimentaire pour non-respect de la signature de la date de signature des conventions, enfin le législateur vient d'adopter, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'application du droit de l'Union européenne, une disposition instituant la possibilité d'associer à une injonction administrative une astreinte financière dissuasive, le gouvernement est donc particulièrement attentifs à l'état des relations entre fournisseurs et distributeurs, notamment dans cette période de négociations commerciales qui font l'objet d'un suivi spécifique des services de la DGCCRF. monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il vous reste 36 secondes pour répondre. Merci madame la présidente, je partage bien entendu votre analyse sur le foisonnement Textuel, mais je ne partage pas votre conclusion sur le fait que on n'aurait pas assez de recul aujourd'hui pour pouvoir analyser les effets de la loi Egalim très concrètement, on voit qu'un certain nombre de producteurs ont du mal à vivre de leur activité, et cela n'est pas normal, on sait bien, il y a, c'est pour les productions que j'ai évoqué tout à l'heure, le lait et la viande bovine notamment, mais ce ne sont pas les seuls et donc là, il importe d'agir et agir cela veut dire trouver d'autres solutions, le gouvernement a mandaté Serge Papin pour analyser cela mais il faudra que cela puisse produire des résultats en tout cas on attend sur le terrain. Merci l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Stéphane Piednoir au secrétaire d'État auprès des ministres de l'Économie et des finances et de la relance et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, à l'heure de la dématérialisation quasi généralisée en France comme ailleurs, l'outil informatique est devenu quasi incontournable pour toutes les tâches du quotidien et pour toutes les tranches d'âges de la population, chacun est de plus en plus inciter à avoir recours à des actes dématérialisé pour pour des, des, des services au quotidien, c'est d'autant plus vrai en période de confinement que nous avons traversée avec le développement du télétravail, bien sûr, mais d'une manière générale, les démarches administratives sont de plus en plus à effectuer en ligne et les commandes passées sur Internet évidemment ont progressé également cet outil constitue bien sûr à bien des égards à un progrès incontestable, son utilisation peut néanmoins s'avérer complexe pour certains utilisateurs au-delà de simples difficultés d'usage de nombreux actes malveillants arnaque piratage peuvent duper les utilisateurs, ce phénomène n'est malheureusement pas nouveau, bien entendu, mais il a connu une forte augmentation depuis le confinement avec notamment l'émergence de sites frauduleux des fausse cagnotte des usurpations d'identité ou encore des escroqueries en tous genres, la recrudescence de ces arnaques sur internet touche pas tout le monde mais impacte tout particulièrement les seniors, souvent, on le sait moins à l'aise avec l'outil informatique, c'est ce que dénonce, par exemple, la Confédération française des retraités de Maine-et-Loire qui entreprend des actions de sensibilisation pour lutter contre la multiplication des arnaques sur internet lors de votre déplacement en Seine-Saint-Denis le le 15 janvier dernier Monsieur le Ministre, vous avez rappelé l'objectif du gouvernement de faire du numérique, un outil au service de tous au service de notre quotidien et de l'émancipation citoyenne dans ce cadre, Monsieur le Ministre quelles actions entendez-vous pour mettre en place pour mieux informer et protéger les utilisateurs d'internet. Merci, la parole est à monsieur Cédric au secrétaire d'État. Oui, madame la la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, vous évoquez ce fléau des attaques sur internet qui se développe de plus en plus, notamment à l'occasion du confinement. Certaines catégories de la population dans les seigneurs moi senior, pardon, moins à l'aise avec les outils numériques peuvent plus facilement être dupés par des arnaques en ligne, toutefois, il serait illusoire de croire qu'un jeune connectés, ne peut pas également être victimes de telles attaques de fait très dépendant du numérique avec d'usage multiple, les jeunes sont également une cible privilégiée des arnaques sur Internet, et force est de constater que nombre d'entre eux se font piéger la réponse du gouvernement face à ce phénomène se décline en 3 volets complémentaires, la sensibilisation, l'assistance aux victimes et la répression en matière de sensibilisation et d'assistance aux victimes, l'action du Groupement d'intérêt public : cybermalveillance Point gouv Point FR doit être souligné, associant des organisations, des associations professionnelles, de grandes entreprises et des services de l'État, ce GIP diffuse largement des conseils en matière de sécurité numérique au profit au profit des particuliers, il réalise des annonces de sensibilisation et des campagnes d'affichage massive dans les Cars, par exemple, certains des membres du GIP réalise également des campagnes de sensibilisation, je reconnais bien volontiers que la sensibilisation des Français aux problématiques de sécurité numérique reste encore trop faible, et nous y travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour sensibiliser les élèves avec le ministère du Travail avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ainsi qu'avec les entreprises du secteur concernant l'assistance aux victimes, la plateforme plateforme cyber malveillances Point gouv Point FR je là aussi un rôle essentiel, elle offre un parcours automatisée extrêmement simple et didactique pour toute personne ayant subi une action Internet ou une cyberattaque au travers de quelques questions, la plateforme oriente les victimes pour qu'elles reprennent le contrôle de leurs équipements dans les cas les plus simple ou qu'elles aient recours aux services d'un professionnel référencés sur la plateforme, lorsque l'atteinte est plus grave, enfin il est indispensable que ces arnaques toutes comme celle perpétrée dans le monde physique ne restent pas impunis à ce titre j'encourage évidemment toutes les victimes de ces arnaques à se rendent dans le commissariat de police ou dans la brigade de gendarmerie la plus proche. Et à porter plainte, trop souvent, celle-ci s'interdisent de le faire, on pense que ce n'est pas utile garde l'attaque pour elle-même, cela nous empêche de poursuivent les auteurs et cela doit conduire à ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui portent plainte afin que nous puissions réprimandé justement les personnes qui se livrent à ces contraventions trop souvent les victimes, je le disais le font trop peu souvent et porte seul ces difficultés, les plaies les plaintes nous permettent et permettent au service d'enquêteurs d'obtenir la vision la plus complète possible des atteintes commises et conduisent de plus en plus fréquemment à des arrestations. Merci, cher collègue, il vous reste une trentaine de secondes pour répondre. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je partage vraiment votre analyse sur le fait que ces ces arnaques peuvent concerner évidemment les les jeunes publics souvent par naïveté les les publics plus avancée en âge, les seniors sont se font avoir, si je puis dire, par des, des, des sites qui sont extrêmement bien fait qui s'apparentent à des sites gouvernementaux, parfois sans doute faudra-t-il davantage les sensibilités sur le dernier point que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité de porter plainte, de porter de de faire en sorte que les sanctions qui soient prononcées contre les auteurs de ces sites frauduleux et je pense que vraiment une sensibilisation directement directement sur les sites pourraient être via des codes pour être instituée très prochainement en tous cas je vous sais impliqué sur ce dossier du numérique merci. Merci, cher collègue, l'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Bruno Roche joint au secrétaire d'État auprès des ministres de l'Économie, des finances et de la relance et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaite vous alerter quant aux problématiques liées à la couverture en téléphonie mobile dans les territoires ruraux, selon les statistiques officielles, la couverture en téléphonie mobile du département de l'Allier est considérée comme bonne 99 % du territoire est couvert, selon l'Arcep, seulement il existe une part non négligeable du département au sein de laquelle cette couverture n'est assurée que par certains opérateurs ainsi dans 17 % du département au moins un des opérateurs est défaillant et n'offre pas de couverture hanté en réseau mobile, la plupart de nos concitoyens n'ont qu'un seul abonnement mobile et se retrouvent avec des trous de couverture lorsque leur domicile et leur lieu de travail n'est pas couvert par le même opérateur ou lorsqu'il se déplace, il est ainsi difficile de mener une vie normale d'accéder aux services de secours de permettre le dynamisme économique des territoires et de les rendre attractif. Cette situation rencontrée dans l'Allier, l'est également dans d'autres départements ruraux, il apparaît donc pertinent qu'un opérateur dès lors qu'il est le seul à couvrir une zone rurale soit obligés d'assurer, via ses propres équipements la couverture pour le compte des autres opérateurs cette pratique appelée Ran sharing permet à des opérateurs d'être présent sur une zone peu rentables sans investissements lourds et d'améliorer significativement la couverture mobile pour ses habitants, je souhaite par ailleurs attirer votre attention sur les mesures de couverture mobile utilisé par l'Arcep comme par les opérateurs, si elles permettent d'afficher des taux de couverture très élevé, elles sont très contestables, dans les faits, ces mesures reposent sur des simulations numériques et se base sur des niveaux de signal théorique en extérieur, dès lors, dans beaucoup de zones considérées comme couverte, il n'est en fait pas possible de capter le réseau mobile à l'intérieur du bâtiment, la situation sur le terrain et donc bien plus dégradée que ce que laissent penser les statistiques aussi, je vous remercie de nous indiquer, Monsieur le Ministre, les intentions du gouvernement quant à la généralisation du sharing et de toute autre initiative visant à améliorer la couverture réseau en milieu rural, ainsi que les actions que compte mener le gouvernement afin de généraliser l'utilisation d'indicateurs fiables, prenant en compte la pénétration à l'intérieur des bâtiments pour évaluer l'étendue de la fracture numérique, qui reste une réalité dans les territoires ruraux. Merci, cher collègue, la parole est au secrétaire d'État Monsieur Cédric O. Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, étions tous les 2, il y a, il y a 3 jours, dans votre département, pour incarner la volonté du gouvernement de s'attaquer de manière extrêmement décidée à cette problématique de la fracture numérique, qu'elle soit d'ailleurs par action numérique par la connexion réseau mobile ou fracture numérique par les usagers, ce qui a conduit le gouvernement à travers notamment le plan de relance, mais aussi un certain nombre d'autres dispositifs, notamment le fameux dispositif New Deal investir des sommes inédite dans la réduction de cette fracture numérique s'agissant de la question vous avez raison, Monsieur le Sénateur, l'impatience de nos concitoyens et légitime et elle existe toujours, le déploiement de nouveaux pylônes et toujours trop lent et toujours trop, je je vais tout de même rappeler les chiffres qui sont ceux du New Deal mobile entre 2003 et 2018 le précédent plan France blanche a conduit les précédents gouvernements à déployer en 15 ans 600 pilotes en zone blanche grâce au New Deal mobile signé en juin 2018 entre juin 2018 et fin 2022, ce seront 2500 pylônes qui seront allumés en zone blanche, nous sommes donc passés d'une dynamique de 600 pilotes dans 15 ans en zone blanche à 2500 pylônes en 2 ans et demi au total ce sont 10 à 12000 pylônes qui seront allumés dans des zones blanches et qui permettront de réduire extrêmement drastiquement la fracture numérique s'agissant du département de l'Allier, j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma récente visite, ce sont 39 nouveaux sites mobiles qui ont été jugés comme prioritaires identifiés par l'équipe projet de l'Allier, ils ont fait l'objet d'un arrêté 6 nouveaux sites mobiles d'ores et déjà été mis en service, ce sont 33 nouveaux sites qui ouvriront d'ici fin 2022 je rappelle également que la méthodologie a changé, il ne s'agit plus de s'appuyer sur des mesures théoriques, comme vous l'avez évoqué mais ce sont les élus locaux avec le préfet du département, qui décide des endroits où seront déployés les pylônes des automobilistes qui nous permet de répondre à la réalité du vécu de nos concitoyens, je rappelle également que le choix est laissé aux territoires de prioriser des zones dites blanches, c'est-à-dire où il n'y a aucun opérateur ou des zones dites grises, c'est-à-dire des zones où un ou plusieurs opérateurs sont présents, ce qui permet une flexibilité pour permettre de s'adapter aux caractéristiques locales lorsqu'une zone dite blanche et prioriser localement les 4 opérateurs sont obligés de mutualiser leurs infrastructures, dans le cas du Ran sharing, que vous avez évoquée lorsqu'une zone d'Itinéris et prioriser le dispositif permet de compléter la couverture avec les opérateurs non présent à ce stade et d'apporter ainsi la couverture de l'ensemble des opérateurs sur le territoire concerné, je conçois que l'impatience de nos concitoyens souhaitent grande mais je veux vous assurer monsieur le sénateur, vous avez eu l'occasion de le voir sur le terrain, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, également, que la mobilisation du gouvernement pour mettre fin aux zones blanches et totale, je vous remercie. monsieur le secrétaire d'État à l'ordre du jour appelle la question orale de Madame Anne Van talons au Ministre de l'Économie, des finances et de la relance. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, le 30 octobre Bruno Le Maire, déclaré le télétravail est la règle, le reste c'est l'exception pour de nombreux habitants de la ruralité et particulièrement en Ardèche cette exception relève de l'ordinaire, particuliers, entreprises, collectivités personnes isolées ou fragiles, tous subissent encore et toujours, les déboires de réseaux filaires obsolète et dysfonctionnel en 2021, un accès à une téléphonie fixe de qualité ne devrait pas être une chance mais un droit garanti, comme l'eau ou l'électricité, hélas, l'entretien désastreux du réseau en cuivre empêche de nombreux abonnés de bénéficier du service universel de téléphonie pour tendu par l'opérateur historique Orange, tandis qu'Orange est tenu d'intervenir en 48 heures, les délais de réparation se compte en semaines et de simples ouverture de ligne réclame des mois ainsi une demande de raccordement de l'dans la commune de l'ironie en Ardèche et datant de n'en n'a pas abouti à ce jour, dernièrement, ce sont les communes ardéchoise, des attaques de Saint Martial et du croc de qui ont eu à subir cette impéritie au sol poteaux tombés réactivité médiocre et délais de traitement de pannes extravagant orange a été désigné en 2017, par le ministre de l'économie pour piloter le contrôle du service avec des indicateurs nationaux et ceci pour une durée de 3 ans en 2018, l'Arcep, constatant qu'Orange de respecter pas ses obligations l'mis en demeure d'apporter les indispensables amélioration sur plusieurs indicateurs notamment les délais de raccordement et d'intervention, faute d'investissements et d'une quelconque volonté de la part d'un opérateur qui misent sur le déploiement de la fibre et de la 5 G aucune amélioration notable n'a été apportée depuis vous avez vous-même déclaré qu'il y avait urgence et missionné une députée à ce sujet, or la convention avec l'État, est arrivé à échéance le 27 novembre 2020, ma question concerne donc le cahier des charges de celle qui doit la remplacer inscrire et vous des critères plus lisible permettant d'apprécier la situation propre à chaque département afin de résorber enfin les problèmes de la téléphonie fixe en milieu rural. Merci, cher collègue, la parole est au secrétaire d'État, Cédric O. Oui, madame la la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous évoquez un problème qui concerne effectivement actuellement beaucoup de nos concitoyens, comme vous l'avez dit le gouvernement, les opérateurs ont un objectif de déploiement de la frime, qui est extrêmement important, qui doit conduire à une forme de service universel d'ici fin 2025 et apporter la fibre à tout le monde dans l'attente, beaucoup de territoires beaucoup de Françaises, Français, dépendent encore du téléphone fixe du réseau cuivre pour pouvoir comme unifiée avec l'extérieur et ce téléphone fixe ce ce réseau qui privé est absolument indispensable pour ce réseau cuivre était régis par un service universel dans la convention avec Orange a pris légalement, enfin le 4 décembre dernier, vous l'avez évoqué nous devions voter dans le courant de l'année précédente, le projet de loi d'adultes transposant la directive européenne qui encadre les conditions du nouveau service universel, compte tenu du Covid vous n'avez plus madame la sénatrice voter ce projet de loi des du que fin décembre et nous sommes en quelque sorte, dans une période de transition où le précédent service universel a pris fin et le nouveau service universel doit être défini les services de l'État, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales travaillent extrêmement dur à la définition de ce nouveau cas de service universel dont il est probable d'ailleurs qui doivent s'adapter à la réalité quotidienne des territoires, mais pour être extrêmement concret ce nouveau cadre prendra probablement plusieurs semaines voire plusieurs mois à être défini, or il est hors de question de laisser nos concitoyens et nos concitoyens qui aujourd'hui sont coupés du téléphone ou bénéficie d'une insuffisante qualité du réseau cuivre sans solution, c'est pourquoi vous l'avez évoqué l'ensemble national a décidé de confier une mission flash, c'est-à-dire d'un mois à la députée Célia de Lavergne, appuyés par les services de mon ministère afin qu'elle puisse faire des propositions au gouvernement, en lien avec les différents acteurs d'ici un mois, un mois et demi afin d'avoir une réponse rapide, rapide, car ce que nous voulons, c'est faire en sorte d'apporter une réponse à l'ensemble des Françaises et des Français qui n'ont pas de solution aujourd'hui dans l'attente de la définition de ce nouveau cadre de service universel, je l'ai dit, vous m'avez cité il y a absolument urgence on doit déployer la fibre on doit déployer le réseau mobile, je le disais tout à l'heure, mais on doit aussi, le temps que la fibre soit généralisée à l'ensemble du territoire et l'ensemble des Français, maintenir une bonne qualité du réseau cuivre. spécifier que je resterai attentive à vos décisions et à vos actions, gardant en tête que, il y a un état d'urgence et que la téléphonie fixe est un droit et le service, la qualité de service à une nécessité merci un devoir Merci, chers collègues, mes chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour l'examen de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, la séance est suspendue.